les propos d'un surveillant pénitentiaire au sujet de Flavien Moreau, premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, libéré avant-hier. Condamné, en 2014, à sept ans d'emprisonnement pour terrorisme, cet homme a été libéré un peu moins d'un an avant la date prévue, malgré une détention parsemée d'incidents. Sa sortie de prison s'accompagne d'une double mesure de surveillance, judiciaire- d'une durée de onze mois et dix-huit jours -et administrative. Son cas n'est pas isolé, puisqu'une quarantaine de djihadistes français ont retrouvé la liberté depuis 2018, et que plusieurs dizaines d'autres devraient être relâchés cette année. Les solutions d'un tribunal international et du maintien des djihadistes français en détention à l'étranger posent question. En effet, le contexte géopolitique de la région et le délitement de certains États ne permettent plus de garantir que les terroristes y soient jugés et maintenus en détention. Faute de solutions, le rapatriement de djihadistes français apparaît de plus en plus comme une hypothèse envisageable, comme vous l'avez récemment rappelé, madame la garde des sceaux. Seulement, cette question du rapatriement des terroristes français et de leur libération soulève le problème de la récidive. Comment s'assurer de l'absence de dangerosité de ces individus une fois libérés ? Madame la garde des sceaux, la lutte contre la radicalisation est un combat de longue haleine. Face à de tels criminels, notre arsenal juridique est insuffisant.

Aujourd'hui, la colère s'étend jusqu'à gagner tous les services hospitaliers. Le 20 novembre dernier, le Gouvernement a présenté son plan d'urgence, articulé autour de trois axes : restaurer l'activité de l'hôpital, déverrouiller le fonctionnement de celui-ci et dégager des moyens supplémentaires.

qui ont démissionné de leurs fonctions administratives pour dénoncer les conditions de travail détériorées, le manque de plus en plus flagrant de moyens et les problèmes de relations et de compréhension avec l'administration. Madame la secrétaire d'État, nous ne pouvons pas, bien sûr, vous faire porter le chapeau en vous rendant totalement responsable de cette situation. La lente détérioration des conditions d'exercice au sein des établissements hospitaliers publics a commencé avec les 35 heures, voilà bien longtemps. Comment pensez-vous pouvoir enrayer cette épidémie et rétablir un lien de confiance entre le personnel hospitalier, l'administration et les autorités sanitaires ? Répondre à cette question me paraît essentiel pour ne pas aggraver une crise des vocations déjà vive

de reconnaître certaines contraintes particulières par le biais de primes, de créer les lits supplémentaires nécessaires et de moderniser les conditions de travail. Ces mesures vont changer concrètement le quotidien des soignants et des patients

propos tenus par le Président de la République le 10 janvier dernier, à l'occasion de la rencontre d'échanges avec les 150 membres de cette convention. Expérience démocratique inédite en France et très regardée par nos voisins européens, la Convention citoyenne pour le climat a pour vocation de donner la parole à des Françaises et des Français tirés au sort, avec le mandat de définir une série de mesures qui permettront d'atteindre une baisse d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, dans un esprit de justice sociale. égard, j'observe qu'une nouvelle étape de la fermeture des centrales à charbon a été franchie, avec la signature des contrats de territoire du Havre, de Saint-Avold et de Cordemais. Chacun s'accorde à admettre que la composition de la Convention reflète la diversité des catégories socioprofessionnelles au sein de notre population. Par ailleurs, une attention très forte a été portée au respect de la parité, ainsi que de la diversité des zones géographiques et des types de territoire- territoires urbains, ruraux ou intermédiaires. Sans conteste, cette diversité est essentielle à la qualité des délibérations des six groupes qui travaillent depuis le mois d'octobre dernier. Le Président de la République a pris l'engagement que leurs propositions législatives et réglementaires seraient soumises, sans filtre, soit à référendum, soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe. Dans une période de défiance vis-à-vis du politique, c'est là une méthode originale, consistant à ouvrir le chemin du politique en décelant des voies de consensus dans la société. Nous mesurons bien, collectivement, que nous sommes à un moment où il est nécessaire de privilégier les voies d'un consensus démocratique. Pour ce faire, la Convention citoyenne, dont les membres sont tirés au sort, peut constituer un levier. Démocraties représentative et participative ne doivent pas être en concurrence ni se regarder en chiens de faïence, mais travailler ensemble pour faire face, notamment, à l'urgence climatique qui s'impose à nous. « Si l'on veut réussir cette aventure démocratique inédite, j'ai besoin que vous sachiez prendre des options fortes », a aussi déclaré le chef de l'État le 10 janvier. Prendre des options fortes, c'est aussi l'apanage de la démocratie représentative. Comment le Gouvernement envisage-t-il l'articulation entre cet exercice inédit de démocratie citoyenne et les représentants de la Nation que nous sommes ?

Pour la démocratie, d'abord, parce que nos concitoyens aspirent à participer de plus en plus à l'élaboration des politiques publiques. C'est, d'une certaine manière, la continuation de la dynamique à l'oeuvre dans le grand débat national. Pour l'écologie, ensuite, parce que nous avons besoin de mesures fortes, qui embarquent tous les Français.

Ces citoyens sont extrêmement soucieux, voire inquiets, de ce que nous ferons de leurs propositions. À cet égard, leur rencontre avec le Président de la République, qui a répondu à leur invitation, a permis de réaffirmer l'importance que nous accordons au travail de cette convention et de confirmer la suite qui lui sera donnée.

République a également pris l'engagement de revenir devant la Convention citoyenne pour préciser les modalités de mise en oeuvre. Les propositions les plus abouties pourront être soumises au référendum ou au Parlement- on voit bien là l'articulation entre ces deux formes de démocratie -ou faire l'objet d'un texte réglementaire. Celles qui sont moins finalisées pourront donner lieu à un travail entre les parlementaires et les citoyens. Enfin, le chef de l'État a exprimé son soutien à l'idée d'un référendum, probablement à questions multiples, pour prolonger ce débat démocratique sur l'écologie. Face à l'urgence climatique, les citoyens sont de plus en plus convaincus qu'il faut agir. Nous allons construire les réponses avec eux pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, monsieur le secrétaire d'État chargé des retraites, on peut adhérer aux grands principes du projet de réforme des retraites : régime universel avec suppression des régimes spéciaux, système à points, équilibre financier. On peut aussi comprendre la nécessité de mesures destinées à assurer, à court et moyen termes, l'équilibre du régime actuel, avec ou sans mesures d'âge. On peut également imaginer utiliser le Fonds de réserve des retraites ou accélérer le rythme de la réforme Touraine sur la durée de cotisation. Bien sûr, il faut aussi prévoir le financement de la phase de transition. Mais, en ce qui concerne la réforme systémique, qui prendra pleinement effet en 2037, donc dans dix-sept ans, je m'interroge sur la compatibilité d'un âge d'équilibre prédéfini avec un système à points. Dans un tel système, on conserve une date à partir de laquelle on peut faire valoir ses droits à la retraite- 62 ans -, et le montant de la pension est calculé en multipliant le nombre de points acquis tout au long de la carrière, avec d'éventuelles bonifications, par la valeur du point. C'est une forme d'individualisation de la retraite. Mettre en place un système par points cotisés fait disparaître la notion de retraite à taux plein et relativise les critères d'âge et de durée de cotisation. Dans ce cadre, l'introduction d'un deuxième âge de référence,

l'âge légal, qui est l'âge à partir duquel on peut faire valoir ses droits à la retraite. L'âge d'équilibre sera, au fond, l'âge de départ à taux plein.

nos concitoyens à travailler- c'est vrai -plus longtemps pour- c'est vrai -équilibrer le système de retraite par répartition. Il n'y a là ni gros mots ni scandale : c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde

tout le monde, mais en créant une incitation qui prendra en compte la réalité des parcours professionnels : non pas l'appartenance à telle ou telle entreprise, à tel ou tel statut, mais bien la réalité du parcours professionnel. Ainsi, la pénibilité,

que des chirurgiens soient contraints d'annuler des interventions sur des enfants quelques minutes avant de commencer ? Que des enfants en urgence pédiatrique soient transférés à des centaines de kilomètres ?

%, d'un arrêt immédiat des fermetures d'établissement, de service et de lit, du recrutement en urgence de 100 000 personnes et de l'augmentation des salaires de toutes les catégories professionnelles-

la refonte en profondeur de notre système de santé. Nous faisons en sorte que la médecine de ville se réorganise, afin que la charge n'incombe pas uniquement

proposons également une refondation en profondeur de l'hôpital public : une plus grande délégation de tâches entre les soignants pour libérer du temps médical, des primes pour mieux reconnaître les carrières et des crédits dédiés ? Permettez-moi de vous apporter quelques éléments spécifiques sur votre région. Dans les Hauts-de-France, cet investissement au quotidien représente aujourd'hui 13,8 millions d'euros. 6,3 millions d'euros, dont292 000 euros pour le centre hospitalier de Douai, 550 000 euros pour le centre hospitalier de Roubaix et 371 000 euros pour le centre hospitalier de Tourcoing. 1,5 milliard d'euros seront aussi débloqués sur trois ans pour augmenter les tarifs hospitaliers, ce qui n'a pas été fait depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la reprise de la dette sera engagée à hauteur de 10 milliards d'euros. S'agissant des ouvertures de lits, Agnès Buzyn a demandé aux hôpitaux de faire remonter leurs besoins en aval des urgences. Elle s'est rendue lundi à Corbeil-Essonnes pour constater le déploiement de ces mesures. Les résultats arrivent. La parole est d'euros d'investissements sur trois ans ne permettra pas à l'hôpital public de se relever. Il faudra bien que le Gouvernement finisse par entendre et respecter la colère, les exigences et l'esprit de responsabilité qui montent dans tout le pays, pour sauver notre hôpital public ou notre système de retraite.

c'est heureux. Je suis convaincu que dénoncer de telles dérives, c'est rendre hommage aux milliers de policiers qui font leur travail difficile et dangereux avec maîtrise et qui nous protègent au sacrifice même de leur vie.

depuis des années face au terrorisme et, depuis plus d'un an, dans le cadre des manifestations de protestation sociale, accomplissent leur mission avec sang-froid et dans le respect de nos principes républicains. Pouvez-vous nous dire si vous pensez, au-delà de la déontologie nécessaire qu'il faut faire respecter, que votre nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, qui avait sonné comme un permis de se lâcher,

Vous ne pouvez pas ignorer, car le phénomène a commencé sous le quinquennat précédent, que nous avons affaire à des manifestations de plus en plus violentes. Souvenez-vous des manifestations contre la loi El Khomri. Nous avons vécu avec les « gilets jaunes » et nous vivons actuellement avec les manifestations contre le projet de réforme des retraites, en raison de l'engagement de certaines mouvances ultra, des actions extrêmement violentes qui visent nos institutions

J'observe que la droite le conteste. Bien entendu, je condamne avec force les casseurs. Rendre hommage aux policiers, c'est condamner les dérives qui ont eu lieu.

à mon tour interroger le Gouvernement sur le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie puis libéré ce lundi de la prison de Condé-sur-Sarthe. Cet individu avait été condamné en novembre 2014 à sept ans de prison fermes. cette première sortie va constituer aux yeux de beaucoup de nos concitoyens un véritable test de notre capacité de suivi et de contrôle des djihadistes rentrés dans notre pays, détenus puis libérés après avoir purgé leur peine.

par un juge spécialisé, ainsi que d'un suivi administratif- elle a cité l'obligation de pointage, l'interdiction de quitter son domicile Premier ministre, que ce dispositif prévu pour des détenus de droit commun suffira à rassurer les Français et à assurer leur sécurité ? A-t-on vraiment les moyens d'être efficace, quand on sait que 20 agents sont nécessaires pour surveiller une personne 24 heures sur 24 ?

Premièrement, les condamnations pénales dont font l'objet les personnes qui sont allées sur les terrains de combat sont des condamnations sévères. Depuis 2015, notamment avec l'ancien procureur François Molins, nous avons criminalisé l'association de malfaiteurs terroriste, afin

Une telle cacophonie démontre que le Gouvernement navigue à vue, et nos concitoyens assistent avec consternation à ce barguignage incessant sans obtenir de réponse fiable quant à cette fameuse réforme des retraites. On ne modifie pas l'un des piliers de notre contrat social sur un coin de table entre deux concertations. Âge pivot, âge d'équilibre, incitation à la capitalisation pour les hauts revenus, et, depuis hier, contrairement aux engagements, possible modification de l'âge légal par voie d'ordonnance : mais de qui se moque-t-on ? Les Français ne sont pas seulement inquiets, monsieur le ministre ; ils désapprouvent votre réforme et soutiennent majoritairement les grévistes, car ils ont compris que tout le monde y perdra. Même le seuil minimal de 1 000 euros que vous vous targuez d'instaurer ne serait accessible que pour une carrière continue au SMIC. Le masque de la bonne gestion et de la justice peine à dissimuler les inégalités profondes que vous vous apprêtez à entériner dans un projet de loi bâclé. Personne n'est dupe : vous rejouez en vérité la réforme de l'assurance chômage en mettant au pied du mur les syndicats. Après avoir sciemment organisé le définancement des régimes au travers d'exonérations de cotisations et du recul de l'emploi public, vous appelez à une conférence des financeurs orchestrée pour aboutir à un désaccord des partenaires sociaux et passer en force par voie d'ordonnance. Vous méprisez enfin le Parlement, qui devra se prononcer dans le cadre de la procédure accélérée sur une réforme tronquée de son financement. Il s'agit là d'un coup de force inédit pour le Parlement. Une majorité de Français vous le demande : quand allez-vous faire preuve de discernement et retirer votre texte au profit d'un véritable dialogue social, le temps de présenter une réforme honnête et juste aux Français et à leurs représentants ? La parole est à M. le Premier ministre.

proposer des mesures, qui, si elles permettent de revenir à l'équilibre et respectent les deux bornes que nous avons fixées et qui ont été admises par les organisations syndicales elles-mêmes-

ma détermination personnelle est justement d'en changer, afin que nous dépensions moins et mieux, que nous réduisions par conséquent la dette Ces propos résonnaient dans l'hémicycle comme une leçon un tantinet provocatrice, voire un tant soit peu arrogante et méprisante. Monsieur le ministre,

la dette est à 100 % du PIB, le déficit public est à 100 milliards d'euros et vous prélevez aux contribuables plus de 1 000 milliards d'euros, soit dix fois 100 milliards.

Est-ce que je me satisfais d'un niveau de dette publique aussi élevé ? La réponse est non. Mais ayez l'honnêteté de reconnaître que nous avons réussi à stabiliser la dette publique française alors qu'elle avait augmenté de 33 points au cours des dix dernières années. Ayez l'honnêteté de reconnaître que grâce à ce gouvernement- vous devriez vous en réjouir parce que je sais que vous êtes attaché à la bonne tenue des finances publiques -, la France est sortie de la procédure pour déficit public excessif dans laquelle elle se trouvait depuis dix ans. Ayez l'honnêteté de reconnaître que nous avons engagé un certain nombre de réductions de la dépense publique en matière d'emplois aidés ou de logement qui nous ont permis d'éviter la dérive des finances publiques. il y a eu une crise sociale majeure à laquelle nous avons voulu répondre. C'est la responsabilité du politique de savoir entendre les messages des Français. Les baisses d'impôts que nous avons engagées, notamment la baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse d'un certain nombre de taxes,

dans les deux années restantes du quinquennat pour stabiliser et baisser la dette publique française. Croyez-moi, nous prendrons les décisions nécessaires, et j'espère que vous nous soutiendrez dans ce sens. Monsieur le ministre, Montesquieu écrivait : « J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. » Les Français ne raisonnent pas de travers. Ils ne sont pas dupes : ils connaissent la réalité désastreuse de nos comptes publics. Ma grand-mère, elle, disait : « Ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes. » À force d'arrogance et de mépris, cela pourrait finir « à la lanterne »

Madame la ministre des armées, d'Indelimane à Chinédogar, la liste des attaques meurtrières de djihadistes contre les forces présentes au Sahel s'allonge, et avec elle, celle des victimes, militaires comme civiles, maliennes comme nigériennes, burkinabè comme françaises. Alors que la situation sécuritaire se dégrade rapidement et que la zone d'affrontement s'étend vers le sud, nous observons avec inquiétude qu'une part croissante de la population locale rejette la présence sur place de nos armées. Il était donc important que le soutien des autorités des pays du G5 Sahel à l'appui de la France dans la lutte militaire contre les terroristes soit réaffirmé de manière forte et claire. À cet égard, l'objectif du sommet de Pau est atteint. Toutefois, de nombreuses questions cruciales pour l'avenir de l'opération Barkhane restent en suspens. Le Président de la République a annoncé l'envoi de 220 soldats français supplémentaires au Sahel en appui des forces déjà déployées. L'effort est important, mais au regard de l'intensité et de l'extension géographique de la menace, ce nombre est-il à la hauteur ? Par ailleurs, la déclaration conjointe adoptée à l'issue du sommet exprime la reconnaissance des signataires à l'égard des États-Unis pour leur appui, et demande clairement leur maintien en Afrique de l'Ouest. Or cette demande découle de rumeurs insistantes quant à un éventuel départ américain. Madame la ministre, à quelle échéance aurons-nous des assurances sur ce point crucial ? En cas de retrait avéré des États-Unis, un soutien européen n'en deviendrait que plus essentiel. Nous saluons donc la présence à Pau de Josep Borrell et de Charles Michel, en espérant qu'elle soit le signe d'un renforcement de l'implication de nos partenaires européens. européens. Madame la ministre, pourriez-vous nous éclairer sur la force Takuba que vous appelez de vos voeux, mais également sur la révision du mandat de la Minusma

de Daech, sème le chaos. Pour aider les forces partenaires à reprendre l'ascendant, le Président de la République a en effet annoncé le déploiement immédiat de 220 soldats supplémentaires, mais vous avez raison, l'opération Barkhane ne peut tout faire à elle seule. C'est donc le collectif qui sera la clé du succès. C'est pourquoi, aux côtés des chefs d'Étatdes pays du G5 Sahel, le Président de la République a annoncé la création d'une coalition pour le Sahel. Il s'agit non pas d'une énième initiative, mais d'une nouvelle organisation sous un commandement conjoint, pour plus de renseignement, plus de coordination et donc plus de réactivité. C'est un tournant qui marque l'engagement renouvelé des pays du G5 Sahel, de la France, mais aussi de nos partenaires. C'est un tournant bienvenu dans la perspective de la constitution prochaine de la force Takuba qui regroupera des forces spéciales européennes, afin d'accompagner et d'entraîner les forces armées locales et de leur permettre de monter en compétence dans la lutte contre le terrorisme. Nous comptons en effet sur le soutien précieux des États-Unis pour la réussite de ce dispositif. Nous échangeonsfréquemment avec Washington, et je serai moi-même en visite dans la capitale américaine d'ici à quelques jours, afin de consolider le dispositif existant. Enfin, monsieur le sénateur, au Sahel comme ailleurs, la solution n'est pas seulement militaire : nous le savons bien, il n'y aura pas de sécurité sans développement.

Les Républicains. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, dans cinq jours commenceront les épreuves communes d'évaluation continue en classe de première, épreuves qui s'inscrivent dans la réforme du baccalauréat que vous avez souhaité mettre en oeuvre. oeuvre. Cette première étape importante dans l'évaluation globale des futurs bacheliers de 2021 suscite chez les lycéens un stress bien légitime et bien compréhensible. Cette nouvelle formule

Certains syndicats enseignants appellent même au boycott de ces épreuves, par le biais d'une grève de la surveillance. Si je ne cautionne évidemment pas cette dérive, car je considère que le sens des responsabilités doit l'emporter, celle-ci révèle une rupture du dialogue entre votre ministère et la communauté éducative. Il faut bien reconnaître l'impréparation, pour ne pas dire l'improvisation, autour de ces épreuves : ouverture tardive de la banque de sujets, difficultés liées à la dématérialisation des copies,

Ces épreuves de contrôle continu ont un sens : celui de faire travailler en continu les élèves. Vous avez parlé de « stress » ; je parlerai pour ma part, tout simplement, de travail en continu, dont l'objectif est justement d'éviter le bachotage et de permettre la hausse du niveau des élèves en France. J'entends certains discours ; ils ne sont pas forcément majoritaires. D'ailleurs, les épreuves ont déjà commencé, dans certains lycées, très tranquillement, sans aucun problème, ni humain ni technique. J'observe- vous avez dit que vous ne le cautionniez pas ;

corrigées sur ordinateur. C'est un progrès aussi pour les élèves, puisqu'ils pourront consulter en temps réel leur copie sur ordinateur. Cette dématérialisation est faite.

Vous appelez souvent de vos voeux la construction d'une école de la confiance- c'est même le titre d'un projet de loi que vous avez défendu : confiance envers les jeunes, envers les professeurs, envers les personnels de direction.

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances. En 2018, la France a attiré 339 projets industriels issus d'investissements étrangers, ce qui la place, en la matière, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Près d'un euro sur cinq investis en Europe l'est dans notre pays Dans ce contexte va se tenir le sommet « Choose France ». La première question que je voudrais vous poser est celle de savoir ce que nous attendons, collectivement, de ce sommet, et ce qu'en attend le Gouvernement. Pour redistribuer la richesse, il faut d'abord la créer. Cela vaut d'ailleurs pour l'assurance chômage, la retraite, les accidents du travail, la politique familiale. Si l'État, les collectivités locales, les établissements publics participent et contribuent à cette création de valeur, ce sont d'abord et avant tout les entreprises de notre pays qui créent la valeur. Les premiers bons résultats doivent nous encourager à poursuivre. La France a trop longtemps souffert d'un déficit de compétitivité, qui se traduisait par un déficit commercial et par un taux de chômage élevé.

à redresser la compétitivité de notre pays. Même si les oppositions- c'est leur droit et c'est leur rôle -ne partagent pas cette opinion, je suis convaincu, moi, qu'une grande partie des textes notamment fiscaux que nous avons adoptés ont contribué à renforcer l'attractivité de la France. Créer de la richesse,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la France est devenue la nation industrielle la plus attractive en Europe. Et je pense que cela devrait réjouir toutes les sénatrices et tous les sénateurs de cette assemblée. La France, pour la première fois depuis dix ans, a créé 12 000 emplois industriels en 2018, et 12 000 emplois industriels en 2019. Tous, ici, nous devrions nous réjouir de voir la France redevenir enfin une grande nation industrielle. Et tout ça n'est pas tombé du ciel sénateur, c'est le fruit de la politique conduite par le Premier ministre, par le Président de la République, avec votre soutien. La baisse de la fiscalité

toutes les filières industrielles pour leur donner plus de cohérence et de puissance. Je vous le dis : nous sommes sur la bonne voie, et nous allons redoubler d'efforts pour inscrire ces résultats dans la durée. Le pacte productif sur lequel nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois doit nous doter d'une industrie puissante et décarbonée. Notre objectif, dans les années qui viennent, est d'ouvrir de nouvelles filières industrielles, de nous placer sur les marchés porteurs, d'investir davantage dans l'innovation et dans les nouvelles technologies, de former plus d'ingénieurs et de faire de la France la première puissance industrielle en Europe. C'est à notre portée, et nous y arriverons

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Mme la ministre des solidarités et de la santé, à l'heure où plus de 1 000 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service, lui ont envoyé une lettre de démission collective pour protester contre le dramatique, désastreux et récurrent manque de moyens de notre hôpital public. Au-delà de ce cri désespéré de nos soignants après des années de souffrances dans leurs services, c'est à un véritable burn-out de tout notre corps hospitalier que nous assistons. Les conditions de travail sont telles qu'elles remettent en cause la qualité des soins et menacent la sécurité des patients. Nos médecins et nos personnels paramédicaux ne sont pas des machines. Ce sont des êtres humains qui consacrent leur vie à soigner et à sauver les autres. Notre hôpital public est en déliquescence ; il souffre et il se meurt, parce qu'il est au bord de l'asphyxie

Seule une vraie réforme en profondeur de notre système de santé pourra sauver notre hôpital public ; cela passe par des décisions immédiates, fortes et courageuses

nous demandez d'organiser une transformation en profondeur de notre système de santé ; c'est ce que fait Mme la ministre ; c'est ce que nous faisons au quotidien. Vous nous demandez de mettre en oeuvre une meilleure répartition du travail et du temps médical ; c'est ce que nous faisons en redonnant du temps médical et en permettant une répartition des tâches

Vous nous demandez de mieux articuler la médecine de ville et le secteur hospitalier ; c'est ce que nous faisons avec le plan Ma Santé 2022.

Madame la secrétaire d'État, je vous ai écoutée. Il faut maintenant passer des déclarations d'intention aux financements, et des financements aux actes, pour sortir de cette impasse avant qu'elle ne se transforme en catastrophe sanitaire nationale, et pour dissiper la méfiance légitime de nos médecins et de nos personnels hospitaliers, qui pèse lourdement sur la santé des Français. Très bien ! La parole est à M. Martial Bourquin, pour le groupe socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, le taux du livret A est aujourd'hui à 0,75 nous apprenons qu'il risque de passer, au 1 février, à 0,5 %. Il avait été gelé sous le précédent quinquennat, pour éviter une baisse. Ma question est simple : restera-t-il une épargne populaire dans notre pays ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bourquin, les Français les plus modestes ont eux aussi besoin de logements sociaux. Et vous savez aussi bien que moi que le logement social est financé par le livret A.

l'État emprunte à 0,1 % à échéance de dix ans. Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne sont négatifs. Si nous voulons que le secteur du logement social puisse construire des dizaines de milliers de logements nouveaux pour les Français les plus modestes, il faut que la ressource du livret A soit la moins coûteuse possible pour

n'est jamais inférieur au niveau de l'inflation. Et j'incite le maximum de Français à faire appel à ce livret d'épargne populaire dont nous garantissons que le taux ne sera jamais, je le répète, inférieur

Mais ils sont 34 % parmi les chômeurs. Quand nous faisons baisser le chômage en France, nous apportons donc la meilleure réponse au problème de la pauvreté dans notre pays.

Vous avez plombé votre quinquennat avec la fin de l'ISF et la double année du CICE. Vous avez opéré un basculement inédit de la fiscalité des plus riches

Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Hilarion Tumi Vendegou, qui fut sénateur de la Nouvelle-Calédonie de 2011 à 2017.

Ainsi, un Français sur quatre est exposé à un risque d'inondation, presque toutes les communes de France ont été frappées par une catastrophe naturelle depuis 1982, la sécheresse et ses dommages diffus sur les constructions concernent la quasi-totalité du territoire national et une grande partie du littoral est menacée par des risques de submersion marine et par l'érosion croissante du trait de côte. Les tempêtes, les orages de grêle, les inondations qui ont eu lieu récemment ont encore illustré de manière tragique la vulnérabilité de notre territoire. Cette exposition aux catastrophes naturelles va s'amplifier dans les prochaines années à cause du dérèglement climatique. Ainsi, les pluies extrêmes augmenteront dans toutes les régions et les vagues de chaleur deviendront plus nombreuses et plus fortes, engendrant tous les deux ou trois ans des sécheresses comparables à celle de 2003. Face à cette situation, le groupe socialiste et républicain, auquel j'appartiens, a demandé, en janvier 2019, la création d'une mission d'information. Après six mois de travaux et une trentaine d'auditions,

force est de constater que le système actuel reste incompréhensible et injuste pour de nombreux sinistrés. Les remontées d'informations émanant du terrain dont nous avons été destinataires dressent un bilan sans appel de ce système opacité de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, inintelligibilité des critères utilisés, manque d'explications sur les motifs des décisions prises, délais d'instruction extrêmement longs, etc. Les griefs retenus par les sinistrés à l'encontre du régime d'indemnisation sont légion et conduisent souvent à une remise en cause de la légitimité des décisions de non-reconnaissance. Il est inacceptable que nos concitoyens, après avoir tout perdu lors d'une catastrophe, n'aient d'autre choix que de s'engager, pendant plusieurs années, dans un véritable « parcours du combattant » pour tenter, souvent en vain, d'obtenir une aide des pouvoirs publics ou des assureurs.

En effet, les particularités du phénomène de retrait-gonflement des argiles, et notamment le décalage entre la sécheresse et l'apparition des fissures, rendent son indemnisation plus complexe. À cela s'ajoute le fait que les critères retenus pour apprécier l'intensité de ces épisodes ne rendent pas compte de la réalité du terrain et n'intègrent pas la fréquence croissante de cet aléa. Ces mêmes critères sont également à l'origine d'inégalités de traitement difficilement justifiables entre des territoires voisins, qui engendrent un vif sentiment d'injustice parmi les sinistrés. J'ajouterai que les techniques de réparation proposées par les experts d'assurance ne sont pas toutes efficaces ; certaines aggravent même la vulnérabilité future des habitations Dans ce contexte, et pour concrétiser certaines recommandations de notre mission d'information, j'ai déposé la proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui. Nous appelons à une modernisation durable du système d'indemnisation des dommages résultant de catastrophes naturelles. Il s'agit de renforcer les droits des assurés et de revaloriser le montant

Je pense notamment à la méthodologie retenue pour qualifier un phénomène de catastrophe naturelle, aux dispositifs de franchise qui pénalisent excessivement certains sinistrés, ou encore aux relations entre les assurés et les assureurs, qu'il convient de clarifier. Un effort global de pédagogie à l'égard des sinistrés est également nécessaire, l'information concernant les critères et les seuils d'intervention du régime Cette proposition de loi, au-delà d'une meilleure indemnisation des sinistrés, prévoit également de renforcer le pouvoir des maires, qui sont en première ligne lorsque survient une catastrophe naturelle. Ils se trouvent souvent isolés, parfois même désemparés, quand ils doivent faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle de leur commune, ou quand leur revient le devoir d'expliquer la situation à leurs administrés et de se faire le relais de décisions ministérielles parfois difficiles à comprendre et à entendre. Nous proposons donc de réformer la composition de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle d'allonger la durée pendant laquelle une demande de reconnaissance peut être formulée ; de permettre aux maires de soumettre une deuxième demande de reconnaissance dès lors qu'ils produisent des données complémentaires ; de créer une cellule départementale de soutien aux maires.

L'un des constats essentiels de notre mission d'information est que ce fonds manque aujourd'hui de marges financières, du fait du plafonnement de ses ressources par l'État. Il manque également de souplesse, du fait de l'existence de dispositifs de sous-plafonnement. Il se trouve en outre qu'il est victime de ponctions régulières sur sa trésorerie, Je le dis : cette situation constitue un vrai dévoiement de la contribution versée par les assurés, dévoiement guidé par des considérations budgétaires de court terme.

Ce déplafonnement des ressources du fonds Barnier est un élément essentiel du dispositif que nous proposons aujourd'hui- je rappelle de nouveau que le rapport a été adopté à l'unanimité par les membres de la mission d'information du Sénat. J'espère donc que les divergences d'approches sur ce sujet ne remettront pas en cause l'ensemble de notre texte. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire concernant cette proposition de loi, qui n'a pas de couleur politique- elle est le fruit d'un travail du Sénat, comme celui-ci sait en faire -, qui s'appuie sur la réalité du terrain, qui est attendue par les citoyens et les élus, et dont j'espère, madame la secrétaire

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, seront, à n'en pas douter, l'un des principaux défis liés au climat de la décennie qui s'ouvre. Cette proposition de loi fait suite aux travaux de la mission d'information, à laquelle j'ai participé, qui a rendu ses conclusions en juillet dernier.

sur les dispositions budgétaires, fiscales et du code des assurances, qui relèvent pleinement de sa compétence. Je tiens, pour commencer, à saluer le travail de grande qualité effectué par la mission d'information sous l'autorité de son président, Michel Vaspart, et de sa rapporteure, Nicole Bonnefoy, dont le rapport a parfaitement mis en exergue les immenses difficultés rencontrées par les sinistrés. De la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à l'indemnisation en passant par la prévention des risques climatiques, les sinistrés sont souvent confrontés à un véritable parcours du combattant. Comme nous l'ont encore rappelé les récentes inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes, lorsqu'une catastrophe naturelle dévaste une résidence principale, ce sont, dans bien des cas, les économies de toute une vie qui disparaissent ; la dimension affective de la catastrophe n'est Ainsi, les objectifs des auteurs de cette proposition de loi sont louables et, surtout, fondés, en ce sens qu'ils visent à assurer une indemnisation juste, à la hauteur du préjudice subi, et à mieux mobiliser les dépenses affectées à la prévention des risques naturels.

Sont-elles opérationnelles, tant pour les sinistrés que pour les assureurs et les pouvoirs publics ? Enfin, leur efficacité est-elle à la hauteur de leur coût pour les finances publiques ? ? L'article 1 de la proposition de loi tend à déplafonner le montant des recettes affectées au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Rappelons que la loi de finances pour 2018 finances pour 2018 a plafonné l'affectation au fonds du prélèvement de 12 % sur les primes « catastrophes naturelles » payées par les assurés à 137 millions d'euros par an.

Pour autant, je considère qu'un déplafonnement pur et simple des recettes qui lui sont affectées n'est pas souhaitable. D'abord, ce déplafonnement relève du domaine exclusif de la loi de finances, car il s'agit d'une disposition affectant le budget général de l'État. Ensuite, compte tenu de la variabilité des dépenses du fonds, il pourrait également conduire à l'accumulation d'une trésorerie, dont résulterait un prélèvement par l'État, comme cela a déjà été le cas par le passé. Je proposerai donc de fixer un nouveau plafond de recettes pour le fonds Barnier

en lui confiant la détermination d'un objectif pluriannuel pour les dépenses du fonds. Tout en partageant les intentions des auteurs s'agissant du pilotage stratégique du fonds, je me dois de rappeler que la définition des missions de ce conseil relève non pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire. Les dispositions proposées sont donc contraires à l'article 41 de la Constitution. le décret du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif a procédé à la fusion du conseil de gestion avec le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, afin de clarifier la gouvernance du fonds. fonds. La fixation d'un objectif pluriannuel de dépenses, quant à elle, ne me paraît pas souhaitable, dès lors que ces dépenses sont difficiles à prévoir plusieurs années à l'avance. À mes yeux, la détermination d'objectifs chiffrés pluriannuels sans prise en compte des besoins, évalués au fur et à mesure, au plus près des territoires, n'est pas à même d'améliorer la performance du fonds. S'agissant de l'article 2, son objectif est de garantir une meilleure indemnisation des assurés à la suite de catastrophes naturelles. Si la commission des finances partage cette ambition, plusieurs réserves substantielles ont été soulevées lors de l'examen du texte la semaine dernière. et même bien travaillé -avec la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, Nelly Tocqueville, afin de trouver des compromis. Par conséquent, nous allons vous présenter des amendements identiques

La volonté d'allonger ce délai ne nous a semblé justifiée que pour l'indemnisation des dommages liés aux épisodes de sécheresse, pour lesquels, en effet, les dégâts causés mettent parfois plusieurs années à se manifester et à être bien expertisés. Dans les autres cas de catastrophes naturelles, il me semble au contraire qu'un délai relativement court encourage une résilience rapide des territoires concernés. Deuxième objectif, une rédaction alternative à la disposition selon laquelle l'indemnisation reçue doit « garantir une réparation pérenne et durable, de nature à permettre un arrêt complet et total des désordres Je proposerai plutôt d'insister sur le fait que les réparations effectuées doivent être proportionnées aux dommages et tenir compte des meilleures techniques existantes.

Troisième objectif, la précision des modalités d'intégration des frais de relogement d'urgence dans le périmètre de la garantie CatNat. Cette précision répond à une réelle demande des sinistrés. Enfin, l'article 3 vise à créer un crédit d'impôt au titre des dépenses supportées pour la prévention des aléas climatiques. Ce crédit d'impôt s'élèverait à 50 % du montant de ces dépenses.

aux effets des catastrophes naturelles, et donc de diminuer le reste à charge des particuliers en cas de survenue d'une telle catastrophe, le crédit d'impôt tel qu'il est proposé serait très coûteux pour le budget général de l'État. Son taux apparaît en effet particulièrement élevé, alors même que ces travaux sont bien souvent très onéreux. Je proposerai donc un amendement visant à le plafonner, afin d'en limiter l'impact budgétaire. Mes chers collègues, je souhaite que cette proposition de loi soit adoptée par le Sénat, en y intégrant, bien entendu, les propositions d'amélioration faites par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Les conséquences directes du changement climatique, ces aléas naturels dont la fréquence et l'intensité augmentent, nous imposent de repenser notre régime de prévention et d'indemnisation des catastrophes naturelles. Rappelons que, d'après une étude de la Caisse centrale de réassurance et de Météo France publiée l'année dernière, le changement climatique provoquera une augmentation de la sinistralité au titre des catastrophes naturelles de 50 % à l'horizon de 2050, ce qui conduira le régime CatNat à être de plus en plus sollicité.

Cette mission a d'abord mis en évidence la nécessité d'investir beaucoup plus que nous ne le faisons aujourd'hui dans des actions de prévention des risques. En permettant une réduction de la sinistralité et, donc, du besoin d'indemnisation, cette tant pour éviter et/ou limiter l'ampleur des catastrophes que pour ménager les comptes publics ! Lors du débat organisé au Sénat sur les conclusions de la mission d'information, la ministre de la transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, a reconnu que l'action face à la multiplication des risques climatiques « passera nécessairement par un rééquilibrage et un renforcement de nos efforts en faveur de la prévention, à laquelle nous consacrons aujourd'hui dix fois moins de moyens qu'à l'indemnisation ».

le privant chaque année de 70 millions d'euros, qui sont détournés de la prévention des risques pour alimenter le budget de l'État ? Cette décision est un non-sens écologique et budgétaire, et j'espère qu'il y sera mis fin rapidement, comme le prévoit la proposition de loi. Quant au régime CatNat, il y a urgence, madame la secrétaire d'État, à le rendre plus efficace, plus protecteur et plus transparent. C'est ce que demandent sinistrés et élus, qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre, et donc à accepter, les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Comment comprendre, en effet, que deux communes voisines confrontées aux mêmes dégâts puissent être placées dans des situations différentes au titre du régime CatNat ? L'opacité de la procédure de reconnaissance et des critères retenus nourrit le sentiment d'injustice éprouvé par de nombreux sinistrés. La mission d'information a également mis en lumière les difficultés particulières que posent les phénomènes de sécheresse, dont les conséquences peuvent se manifester avec retard et pour lesquels les prises en charge proposées aux personnes sinistrées peuvent se révéler inefficaces et insuffisantes. Rappelons, là aussi, que plus de 4 millions de maisons individuelles sont construites sur des sous-sols argileux et sont donc très exposées à des mouvements de terrain liés aux phénomènes de sécheresse. Face à cette situation, il n'est pas responsable d'apporter des réponses ponctuelles et partielles, comme l'a fait l'Assemblée nationale en adoptant, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, un amendement du Gouvernement mettant en place un dispositif de soutien exceptionnel de 10 millions d'euros aux victimes aux victimes de la vallée de la Lys affectées par un épisode de sécheresse en 2018. C'est une démarche totalement irrespectueuse des autres sinistrés et du travail des élus, sans compter qu'elle rompt le principe d'égalité Il convient au contraire d'apporter une réponse globale, en réformant le régime CatNat pour mieux tenir compte des phénomènes de sécheresse. Plusieurs amendements que je vous présenterai tout à l'heure Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable partage la philosophie qui inspire les dispositions de cette proposition de loi. Nous avons travaillé en lien avec le rapporteur de la commission des finances, Jean-François Husson, que je remercie de sa disponibilité, ce qui se traduit par le dépôt d'amendements identiques sur un certain nombre de sujets. Cela montre aussi que nous partageons, au Sénat, la même préoccupation d'adapter notre droit aux conséquences du changement climatique. La parole

madame la sénatrice Nicole Bonnefoy, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de m'accueillir cet après-midi pour examiner cette proposition de loi portant sur un sujet important pour le Gouvernement, car il concerne nombre de nos concitoyens. Notre régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a fait ses preuves, mais doit être adapté à l'évolution des risques. Avec l'accélération du changement climatique, nous affrontons une recrudescence des risques majeurs, qui font peser une menace croissante sur nos concitoyens et sur nos entreprises. Nous l'avons observé depuis le début du quinquennat : avec l'ouragan Irma, les inondations dans l'Aude, la canicule ayant sévi cet été ou, plus récemment encore, les inondations dans le Var, notre pays est confronté de plus en plus fréquemment à des épisodes naturels d'une intensité extrême, qui suscitent des dégâts très importants. Dans ce contexte, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles apparaît comme un régime de solidarité unique au monde, mobilisant l'État, les collectivités et les assureurs au service des sinistrés.

1 milliard d'euros par an, dont 550 millions d'euros au titre des inondations et 400 millions d'euros au titre de la sécheresse. Ce sont environ 3 300 reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle par an, au bénéfice de millions de sinistrés sur la quasi-totalité du territoire français. Mais, les événements des derniers mois l'ont prouvé, nous devons faire mieux. Le changement climatique n'attend pas. La France doit être aux côtés de celles et ceux qui, en un battement de cils, ont parfois tout perdu : leur maison, leurs espoirs, leurs économies et, parfois, leurs proches. C'est pourquoi une réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est aujourd'hui nécessaire. Il nous faut un régime moderne, adapté aux enjeux du changement climatique et à l'accroissement des catastrophes naturelles que ce À l'horizon de 2050, le coût des catastrophes naturelles pourrait augmenter de 50 % du fait de l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements, de l'élévation du niveau de la mer et de la concentration des populations dans les zones à risques. Certains territoires, cela a été souligné, seront plus fortement exposés aux risques naturels en raison des dynamiques démographiques et des effets du changement climatique. C'est notamment le cas des territoires ultramarins, avec une forte augmentation de la fréquence des cyclones.

La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et d'indemnisation doit donc évoluer pour être plus simple, plus transparente, plus réactive et plus efficace. Il nous semble également important que ce régime incite davantage à la prévention et contribue à établir une véritable culture de gestion des risques. Vous vous souvenez que le Président de la République, à la suite du cyclone Irma, avait appelé de ses voeux une réforme de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Je me réjouis que ce souhait soit partagé par une coalition aussi large dans cet hémicycle. et l'excellent rapport rendu par Mme la sénatrice Nicole Bonnefoy constituent une première contribution importante à ces travaux. Je me félicite donc de ce texte, dont les principes directeurs sont, à bien des égards, proches des convictions

rapide et complète des sinistrés, comme l'a demandé le Président de la République. Enfin, nous devons penser aux élus locaux et aux maires. Ils sont en première ligne lors d'une catastrophe naturelle. Ce sont eux, en liaison avec les préfets, qui décident des premières mesures d'accompagnement des sinistrés. Ce sont eux qui, une fois le sinistre passé, engagent la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Il faut leur donner les moyens d'agir sereinement et efficacement. Toutefois, les mesures contenues dans cette proposition de loi soulèvent des interrogations techniques. Certaines vont dans la bonne direction, mais d'autres pourraient être retravaillées. S'agissant de l'article 1, nous partageons l'ambition d'une mobilisation dans les meilleures conditions du fonds Barnier pour financer des projets concourant à la prévention des sinistres et à la réduction des vulnérabilités. Il faut évidemment que les moyens engagés soient à la hauteur des besoins. Toutefois, un certain nombre de dispositions sur le fonds Barnier présentées ici, en particulier la question de son plafonnement, relèvent de la loi de finances.

S'agissant des modalités d'indemnisation assurantielle évoquées à l'article 2, le Gouvernement est prêt à travailler sur la question du relogement, sous réserve de consultations supplémentaires visant à en définir les conditions. Nous sommes réservés sur l'allongement du délai biennal de prescription pour la garantie catastrophe naturelle, allongement susceptible de créer de la confusion chez les assurés sans répondre à leurs problèmes les plus urgents. L'introduction d'un principe de « réparation pérenne et durable » ne nous semble pas conforme au principe d'une indemnité proportionnelle au dommage à la base de l'assurance. La création d'un nouveau crédit d'impôt prévue à l'article 3 semble prématurée, alors que plusieurs dispositifs, tels que le fonds Barnier et certaines réductions d'impôt accordées par ailleurs, apportent déjà des réponses concrètes. En matière de procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle évoquée à l'article 4, le Gouvernement partage les objectifs de transparence et d'efficacité évoqués dans le texte. Dans ce but, il a déjà mis en oeuvre des améliorations très concrètes : par exemple, la création d'une procédure de reconnaissance accélérée ou la dématérialisation engagée de la procédure de reconnaissance, via l'application iCatNat, qui permet aujourd'hui à toutes les communes de France de déposer leur demande de reconnaissance par internet en quelques minutes. Nous sommes favorables à une amélioration de la transparence sur les motivations des décisions, tout en veillant toutefois à ne pas alourdir à l'excès les procédures administratives. Enfin, à l'article 5, l'idée générale d'organisation de cellules de soutien aux maires confrontés aux effets d'une catastrophe, cellules d'élus locaux et de personnes qualifiées, est intéressante. Mais elle doit être approfondie, afin de bien coordonner l'action des différents intervenants sur cette matière. Nous proposons donc de pousser plus loin le travail technique sur ces différents points pour parvenir à un dispositif techniquement abouti, et nous ne serons pas en mesure de donner un avis favorable, à ce stade, à la rédaction retenue pour ces mesures. Le Gouvernement s'engage toutefois à approfondir rapidement les travaux et à enrichir le texte en cours de navette parlementaire. Nous lancerons à cet effet une concertation à brève échéance. En effet, au-delà des interrogations techniques que j'ai mentionnées sur plusieurs dispositions figurant dans la proposition de loi, un certain nombre de points me semblent mériter de plus amples consultations avec l'ensemble des parties prenantes. Nous mènerons ce travail dans les prochaines semaines, en nous appuyant notamment sur le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, dont un grand nombre d'élus font partie. J'identifie quatre thématiques principales que nous souhaitons approfondir dans les prochaines semaines. première thématique est l'amélioration du système de franchises, afin de s'assurer d'un traitement équitable de tous les assurés et d'adapter la prise en charge à leur situation : entreprises, particuliers ou encore collectivités. deuxième thématique est l'amélioration de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, pour faire en sorte que ce régime soit mieux connu et mieux compris par les collectivités et par les assurés, en répondant aux exigences de transparence, de rapidité et d'efficacité. La troisième thématique est le renforcement de nos outils de prévention, non seulement en modernisant le fonctionnement du fonds Barnier, mais également en incitant l'ensemble des acteurs, particuliers comme assureurs, à davantage investir dans les mesures de prévention. La quatrième thématique est l'amélioration de la couverture outre-mer. En moyenne, seuls 50 % des biens ultramarins sont couverts par une assurance dommages contre 98 % en métropole. Le Gouvernement a donc lancé une réflexion relative à la résorption du phénomène de non-assurance ou de sous-assurance outre-mer.

Il est dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens que nous parvenions rapidement à des améliorations concrètes et utiles. Il y va, aussi, de l'intérêt du modèle français de solidarité. Dans la suite

plaisir de participer. Je salue d'ailleurs les travaux de mes collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart. Je les remercie, au passage, d'avoir intégré dans leurs conclusions un certain nombre des remarques et propositions de mon groupe et d'avoir réussi à élaborer un rapport approuvé à l'unanimité. Le dérèglement climatique, contre lequel la France et le monde luttent très peu, entraînera une multiplication et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Des cyclones aux méga-feux, des inondations aux sécheresses, personne n'est épargné Cet enjeu de protection des biens et des populations est prégnant, comme l'a souligné la mission : en France, plus d'une personne sur quatre est aujourd'hui concernée. Cette proposition de loi vient donc utilement compléter un système assurantiel à bout de souffle, comme le démontre le phénomène, déjà évoqué, de rétractation-gonflement des sols argileux sous l'impact de la chaleur, dont les conséquences sur des milliers d'habitations sont désastreuses.

l'impératif de lutter à la source contre les causes et les conséquences du changement climatique. Il nous faut, à la fois, changer notre modèle économique de production et nous adapter aux conséquences immédiates du dérèglement, comme nous y invitait notamment le rapport de nos collègues Ronan Dantec et cela en renforçant les normes d'urbanisme et de construction, en économisant la ressource en eau, en améliorant la gestion des cours d'eau, en végétalisant les zones urbaines pour atténuer un peu les effets des canicules, etc. Il faut Il faut renforcer la résilience de nos territoires. Les pouvoirs publics doivent les accompagner, notamment par la mise à disposition d'ingénierie publique, aujourd'hui largement insuffisante. Alors que l'État est censé garantir la sécurité des personnes et des biens contre les éléments naturels, il est aujourd'hui évident que ce sont les collectivités qui l'aident à s'acquitter tant bien que mal de ses missions, et non l'inverse. C'est problématique quand on sait la disette financière touchant lesdites collectivités À ce titre, nous partageons l'idée, défendue aux articles 4 et 5 de ce texte, de renforcer l'information et l'accompagnement des élus locaux, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de l'état de catastrophe naturelle. Sur le fond même de cette proposition de loi, qui souligne l'absence de moyens pour répondre à l'ampleur des phénomènes, nous jugeons nécessaire de revoir le fonctionnement du fonds Barnier et son financement pour le ramener à la hauteur des besoins. Nous partageons donc pleinement l'objectif de l'article 1, tendant à supprimer le plafond mordant instauré en loi de finances, privant le fonds de 70 millions d'euros. Il est bon d'ailleurs de rappeler, cela a été fait, que ce fonds est financé par les assurés à hauteur de 12 % sur l'assurance habitation, et selon les principes de solidarité.

que ces derniers sont difficilement contrôlables d'un point de vue financier. Pourquoi ne pas avoir préconisé, à l'image de l'évolution du CITE, justement, des aides plus directes pour encourager les particuliers à réaliser les travaux prescrits ? Sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, nous défendons l'idée qu'il convient de créer un conseil national, en remplacement de la commission interministérielle. En effet, les accusations de manque de transparence sont fondées et justifient une évolution plus ambitieuse que celle qui est esquissée dans cette proposition de loi.

Ainsi, les préconisations de la proposition de loi à ce sujet nous semblent timides. En particulier, dans le cadre de la création d'une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles, il semble nécessaire de prévoir la présence de représentants de l'État au sein de cette cellule, comme le propose d'ailleurs la rapporteure de la commission de l'aménagement du Enfin, comme nous le proposions dans notre contribution au rapport, nous invitons le Gouvernement à reconnaître les phénomènes de grêle d'une intensité exceptionnelle des catastrophes naturelles et des calamités agricoles. Comme dans le cas du vent, au-delà d'une certaine intensité, il convient que la puissance publique vienne épauler le système privé inadapté. Aujourd'hui, pour nombre de nos concitoyens, notamment les agriculteurs, l'assurance tempête, grêle, neige est beaucoup trop onéreuse. Ils ne peuvent y souscrire et s'exposent à tout perdre. Avec les violents orages que nous avons connus cet été, notamment en Drôme et en Isère, le coût des assurances privées risque de grimper, entraînant un cercle vicieux délétère. Le ministre de l'agriculture avait d'ailleurs promis un groupe de travail pour remettre à plat tout le système assurantiel relatif à la grêle. Sept mois après, nous n'avons aucune nouvelle. Madame la secrétaire d'État, où en est-on ? Il est en est-on ? Il est urgent d'agir ! À ce titre, nous regrettons le rejet de notre amendement sur le sujet par la commission des finances, qui, comme souvent, nous propose une interprétation extensive, voire abusive, de l'article 40

une bonne proposition de loi, tirée des conclusions d'un rapport d'information fouillé et précis, une réflexion menée en bonne intelligence entre deux commissions pour amender substantiellement le texte, et ce sans le dénaturer. Surtout, le texte que nous examinons aujourd'hui articule bien la réflexion globale sur le dérèglement climatique, d'une part, et l'action locale dans l'intérêt des territoires, d'autre part. C'est à l'honneur de notre assemblée. Le crédit en revient aux auteurs de la proposition de loi. Nous travaillons là, de façon concrète et opérationnelle, dans la bonne direction. En un mot comme en cent, le Sénat est aujourd'hui parfaitement dans son rôle, et je tenais à le saluer. C'est un fait avéré, le dérèglement climatique est à l'oeuvre partout. Notre maison brûle. Cette réalité est désormais visible, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle. Nous avons tous entendu la petite musique qui sonnait à nos oreilles ces dernières années. Elle nous avertissait des catastrophes à venir. Nous y avons tous prêté plus ou moins d'attention. Les plus engagés d'entre nous ont même déjà modifié leurs comportements individuels. Mais, jusqu'à très récemment, les discours sur le dérèglement climatique se conjuguaient au futur. Nous devons désormais les conjuguer au présent. Californie, Amazonie, Australie, autant de noms exotiques qui rimaient hier encore avec soleil et chaleur. Ils riment aujourd'hui avec incendies. Les évoquer doit nous obliger à considérer que nul endroit sur la Terre ne sera épargné par le dérèglement climatique. L'erreur consisterait à penser que notre pays n'en souffrira pas. Notre groupe avait d'ailleurs demandé au Gouvernement, en mai dernier, des précisions concernant les critères de reconnaissance de l'état À la vérité, nos territoires sont déjà affectés par le changement climatique et ses conséquences- nous le savons tous ici, nous qui sommes les porte-voix des élus locaux. C'est le cas des Hauts-de-France, qui ont connu ces dernières années des épisodes répétés de sécheresse aux conséquences dramatiques. On pourrait multiplier à l'envi les exemples, chacun de nous en connaît dans son propre territoire. Cela n'a pas échappé aux assureurs qui ont adapté leurs pratiques en conséquence. Pour eux, l'équation est simple : la couverture du risque se fonde sur le produit d'une probabilité et de l'évaluation de dégâts potentiels. Lorsque la probabilité des épisodes climatiques augmente en même temps que l'ampleur des dégâts potentiels- en clair, lorsque les catastrophes naturelles deviennent à la fois plus fréquentes et plus puissantes -, la couverture du risque augmente aussi. Nul besoin de bien connaître la mathématique pour le comprendre ! Assurer un monde climatiquement déréglé est donc plus onéreux. Et ce coût ne peut être supporté que par la collectivité, puisque le climat est aveugle : il frappe les collectivités humaines au hasard, et non à proportion des gaz à effet de serre qu'elles émettent. C'est notre fardeau à tous ; il nous oblige à la solidarité. est la raison d'être du fonds de prévention des risques naturels majeurs, plus connu sous le nom de fonds Barnier. Son clairvoyant instigateur avait déjà compris la nécessité de mutualiser les moyens d'action. Les ressources de ce fonds sont dynamiques, parce qu'assises sur les dépenses assurantielles. Et puisque, dans le même temps, les dépenses liées aux catastrophes naturelles augmentent aussi, c'est le budget dans sa globalité qui enfle. Je partage donc la volonté des auteurs de la proposition de loi de déplafonner les ressources de ce fonds. Rappelons qu'elles sont payées par les assurés, et donc les contribuables. Elles n'ont pas vocation à combler les déficits de l'État et pallier l'incurie budgétaire. Il faut donc augmenter les ressources de ce fonds, d'une part, et réduire les dépenses publiques, d'autre part. Dette climatique, dette publique, même combat Je m'en remets à la sagesse de la commission des finances pour déterminer le meilleur moyen de procéder à ce déplafonnement. Il nous faudra notamment composer avec le « corsetage » budgétaire qui bride trop souvent le travail et les initiatives parlementaires. Il en va de même concernant le crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques. L'idée est assurément bonne. Il faut désormais s'assurer que le mécanisme retenu sera suffisamment attractif et opérant pour que les particuliers s'en emparent sur l'ensemble du territoire. Pour conclure, mes chers collègues, je saluerai enfin la place que le texte accorde aux élus locaux en tant qu'acteurs incontournables d'une politique ambitieuse de prévention des risques climatiques. Les mesures d'accompagnement prévues par le texte répondent utilement aux attentes du terrain. Bien souvent, les élus locaux se retrouvent désemparés face à des catastrophes naturelles, et l'État ne répond pas toujours présent, ou pas assez vite. Or ce sont bien les élus locaux qui connaissent nos territoires dans toutes leurs particularités. Ils sont les mieux à même d'apporter au plus vite les réponses adaptées aux réalités du terrain. Vous l'aurez compris,

Malgré l'expérience des « anciens », ce phénomène a surpris tout le monde et, dans le froid et la nuit, il a fallu en catastrophe éviter, tout simplement, qu'il y ait mort d'homme. Dès le retour de la rivière dans son lit, quelle expérience terrible ce fut que de faire le tour des maisons pour constater les dégâts, crainte pour l'avenir des bâtiments, les difficultés immédiates de mobilité du fait des véhicules perdus, l'épuisement, le froid, l'humidité ! Et puis l'intime, l'irréparable : cette vieille dame hébétée, qui ne se remettra pas d'avoir perdu ses photos de famille, ou cette petite fille désolée pour son cartable. L'équipe des élus, outre son aide concrète au nettoyage et au pompage, doit dans ces circonstances faire preuve d'une extrême réactivité, car elle est coincée en quelque sorte dans cette position inconfortable d'intermédiaire qui doit donner très vite le conseil- et le bon ! -et faire simultanément les déclarations qui lui incombent comme collectivité territoriale, et bien souvent également comme sinistrée. Pour ma part, j'ai été en tout premier auditionnée par la gendarmerie afin de savoir dans quelle mesure la responsabilité du maire pouvait être engagée dans le phénomène de débordement du cours d'eau. Avais-je bien informé les riverains sur leurs obligations ? Existait-il des embâcles dont j'aurais été responsable ? Cet élément de procédure, à savoir identifier les responsables alors même que tout le monde pompait, Dans ces moments critiques, les élus doivent être solides. Ils ont besoin d'aide, pas de tracasseries, face à l'urgence et au désespoir des sinistrés. Il y a quelques mois, alors que je n'étais plus maire, mais sénateur, j'ai été sollicitée par une association très active de sinistrés de la sécheresse. Les échanges avec les victimes m'ont ramenée au souvenir des inondations : phénomène extrême dans le temps rapide ou le temps long, excès ou manque d'eau. Les désordres prennent des voies différentes, mais le résultat est le même, à savoir traumatisme, désarroi, lourdeur administrative, et l'impression qu'on n'arrivera pas à sortir de la catastrophe naturelle, parce que tout est trop long, trop injuste et trop compliqué. Les associations sont un relais important, car elles ont acquis une expertise et permettent de combattre le sentiment de solitude. Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart se sont saisis de ce problème, menant énergiquement une mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation. La proposition de loi que nous étudions ce jour est la suite logique de ses travaux, car elle prévoit de sécuriser administrés et collectivités. Il est grand temps d'introduire plus d'humanité dans ce dossier. La présence d'élus locaux au sein de la commission interministérielle dont relève la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la création d'une cellule de soutien départementale pour les maires concernés, la possibilité pour eux de déposer une seconde demande de reconnaissance si la première a été rejetée, des délais élargis, etc. : voilà des bouffées d'oxygène indispensables dans des procédures au bord de l'asphyxie.

citer le cas des biens communaux non assurables- par exemple le cimetière -endommagés dans des circonstances, comme le coup de vent, ne relevant pas d'une procédure CatNat. Il y a donc des trous dans la raquette ! Veillons ensemble, avec la bienveillance de l'administration, à les combler au lieu de nous y perdre. J'espère, madame la secrétaire d'État, que vous pourrez me répondre sur ces points. Pour les sinistrés, il faut aussi remédier à certaines lourdeurs, de toute urgence ! Je profite de cette intervention pour signaler que j'avais déposé un amendement pour que les sinistrés disposent d'un délai élargi pour faire leurs déclarations. Cet amendement a été largement cosigné, mais ma proposition relevait, semble-t-il, d'une mesure réglementaire ; je l'ai donc retiré. Le Gouvernement est-il prêt à donner une suite favorable à cette demande émanant de nombreuses associations de défense des sinistrés ... Bien sûr ! ... qui, dans certains cas de force majeure- ils sont parfois évacués -, n'ont pas la possibilité de respecter des délais trop contraints ? L'article 2 allonge le délai de prescription et intègre les frais de relogement d'urgence dans le périmètre de la garantie ; c'est indispensable. La proposition de loi insiste sur le volet de la prévention, ce qui relève de l'élémentaire bon sens, de même que la pérennité des réparations. Plutôt que d'aller vers des franchises vécues comme de cruelles injustices, à l'instar de celle qui concerne le défaut de plan de prévention communal, mesure qui ne relève pas de la responsabilité des assurés et met les élus en défaut, ne faut-il pas, par exemple, être plus exigeant sur les études de sol avant construction ? Elles sont certes obligatoires, mais ne font l'objet d'aucune forme de pénalité, si bien que celui qui souhaite faire construire peut être tenté de faire l'économie de l'étude, et ne pas savoir se protéger de ces phénomènes de retrait-gonflement des argiles, qui occasionnent désormais tant de dégâts ? Si plusieurs mesures n'ont aucun impact financier, les articles 1 et 3 traitent néanmoins le sujet des moyens budgétaires dont il faut se doter, même si, devant la multiplication des phénomènes extrêmes, on peut craindre de voir exploser les dépenses d'une façon qui pourrait ne plus être contrôlée ni supportable. Le fonds Barnier, fonds de prévention des risques naturels majeurs, est actuellement plafonné. Or force est de constater que ce principe de plafonnement s'oppose à la montée en puissance des politiques de prévention. Porter ce fond à 200 millions d'euros, tout en le maintenant dans une enveloppe contrôlée, mais libérée du verrou des sous-plafonds, nous semble une position tout à fait équilibrée. De même, la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt, même encadré, ouvre des perspectives extrêmement intéressantes, qui nous conviennent. Les questions assurantielles sous-tendent l'ensemble du dossier, et je voudrais brièvement évoquer certaines des problématiques qui se posent notamment pour l'agriculture. La solidarité nationale doit venir au secours des agriculteurs non assurés, discriminant en quelque sorte ceux qui ont fait l'investissement de l'assurance et qui peuvent se demander pourquoi ils ont payé. Pour éviter cette situation, les politiques publiques incitent les agriculteurs à s'assurer, ce qui ne fait pas forcément le jeu des assureurs qui, de leur côté, sur les années extrêmes successives, voient l'équilibre du système remis en question. Si les extrêmes deviennent la norme, alors, pour une production agricole, quelle sera l'année de référence ? si les mauvaises années s'enchaînent, la référence est si basse que l'indemnisation ridicule est vécue comme une double peine. Finalement, la prise en charge d'un risque presque certain n'est plus une assurance, c'est un service. C'est ce qui arrive lorsque l'aléa devient systématique. Alors que faire quand se profile un risque d'explosion du système assurantiel ? Voilà, madame la secrétaire d'État, les éléments qui ont alimenté nos réflexions. Pour conclure, puisque nous sommes tous concernés, que nous sommes tous des sinistrés en puissance, qu'il y a un vrai enjeu de prévention, de solidarité nationale, de coordination de tous les acteurs, de stratégie et de résilience collectives, que nous avons tous changé notre regard sur les catastrophes naturelles et que nous avons décidé d'agir, le groupe centriste votera pour ce texte. La parole

Ils montrent que la Haute Assemblée prend cette question très au sérieux en étant à l'écoute d'élus locaux en quête de nouvelles solutions face à des catastrophes toujours plus nombreuses et désastreuses. Je tiens à saluer le président de la mission d'information et sa rapporteure, qui ont été les garants du consensus qui a guidé nos débats tout au long des travaux de la mission dont l'aboutissement est cette proposition de loi. Notre réflexion part d'un constat clair et partagé : le régime actuel d'indemnisation mis en place en 1982 a fait son temps. Les catastrophes climatiques se multiplient en France métropolitaine comme ultramarine, avec toujours le même résultat, une trop faible prévention et une trop grande responsabilité pour des élus en plein désarroi. Aussi, les propositions formulées par la mission d'information, si elles n'avaient pas toutes vocation à s'insérer proposition de loi, apportent une réponse complète aux demandes formulées depuis de nombreuses années. L'article 1 de cette proposition de loi vient réformer un fonds Barnier aujourd'hui trop limité pour les défis qui attendent les élus locaux. La suppression du plafonnement des ressources et du sous-plafonnement par actions permettrait de couvrir des dépenses exceptionnelles, mais également d'élargir le fonds au financement des études et travaux de réduction de vulnérabilité en faveur des particuliers. Celles-ci sont aujourd'hui seulement réservées aux travaux prescrits par un plan de prévention des risques naturels. Nul doute que ces dispositions permettraient, d'un point de vue financier, une meilleure prévention des risques à l'échelle de nos territoires. Il semblerait qu'un relèvement du plafond à 200 millions d'euros soit préféré à sa suppression. Nous nous en contenterons, mais avec de sérieux doutes.

Autant dire que le recours à ces outils s'apparente parfois à un parcours du combattant et que leurs utilisateurs sont souvent rattrapés par les événements eux-mêmes. Ainsi, des collectivités qui ont déjà été touchées sont d'autant plus exposées aux risques, et c'est un véritable cercle vicieux qui s'installe. On est, hélas ! bien loin de la logique initiale de gestion de l'aléa et de la réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires, bien au contraire ! Cela a déjà été très bien dit, mais j'y insiste, un renforcement de la prévention ne sera effectif que lorsque les indemnisations seront plus rapides et vice versa. Lorsqu'un Français sur quatre est exposé au débordement d'un cours d'eau, que 25 % des communes ont subi un aléa climatique en 2018, le temps n'est plus à la réflexion, mais à l'action L'instauration, à l'article 2, d'une obligation de réparation pérenne et durable des assureurs et l'allongement du délai de prescription partent d'une bonne intention. Mais je suis consciente de l'absence de portée normative relevée par la commission pour la première mesure, ainsi que du risque de différenciation de la procédure d'indemnisation en fonction de la cause du dommage. L'inclusion des frais de relogement des sinistrés dans le périmètre des garanties CatNat est une évidence, tant elle était réclamée par les sinistrés et les assureurs. J'en viens à l'article 3. Une des clés pour améliorer la prévention est le développement de la culture du risque chez nos concitoyens. Ils doivent, demain, devenir acteurs dans ce domaine. Le décret du 5 décembre 2019 est en ce sens une belle avancée. Il permet que les propriétaires de logements situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) puissent bénéficier d'une subvention allant jusqu'à 80 % des travaux dans le cadre du fonds Barnier. Je suis d'accord avec l'objectif de nos collègues qui vise à aller plus loin avec la création d'un crédit d'impôt. Certes, il sera très coûteux, mais parce qu'il touche directement les Français, il peut être un véritable outil de sensibilisation et d'implication de nos concitoyens dans la prévention des risques. Concernant l'article 4, j'étais et je reste très favorable aux mesures venant lever l'opacité et la complexité de la procédure de classement en catastrophe climatique. À cela s'ajoute le délai de dix-huit mois parfois trop court pour des communes ne disposant pas forcément des moyens techniques en vue de constituer des dossiers de demande aussi rapidement. Je me réjouis donc des mesures instaurant la publicité de l'avis rendu par la commission interministérielle et des rapports d'expertise rendus. Couplées à l'allongement du délai pour présenter une nouvelle demande de reconnaissance en cas de refus, ces dispositions viendront répondre à l'incompréhension de nombreux élus et citoyens, parfois surpris par des décisions violentes prises de manière verticale. Je conclurai mon propos en insistant sur la nécessaire entraide et coopération entre élus locaux lorsque surgissent ces phénomènes. La création d'un véritable réseau permettant la diffusion des bonnes pratiques ne viendra sûrement pas répondre à toutes les catastrophes, mais elle pourra en éviter et en atténuer certaines. Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE, qui est attaché à ces questions, votera bien entendu cette proposition de loi. La parole

nous débattons aujourd'hui d'un sujet que nos collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart connaissent bien, cette proposition de loi reprenant nombre de pistes avancées par la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et le rapport qui s'en est ensuivi, adopté à l'unanimité par notre assemblée. Je ne peux évidemment que saluer, comme mes collègues l'ont fait, le sérieux et le travail de cette mission d'information, travail qui s'est prolongé jusqu'à cette proposition de loi. J'y associe la commission des finances qui a apporté une expertise complémentaire. Au terme des travaux de la mission d'information, il est apparu urgent de changer la politique publique relative aux catastrophes naturelles sur deux axes. La priorité est le renforcement de la politique de prévention, puisque, et cela a été rappelé, 1 euro investi dans la prévision permet d'économiser 7 euros d'indemnisation. politique de prévention, le fonds Barnier aurait un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Par ailleurs, le rapport de la mission d'information conclut sur la nécessité de réformer le régime des catastrophes naturelles.

De nombreux particuliers signalent des difficultés avec les assureurs lors de la phase d'indemnisation, notamment en matière de délais de déclaration des sinistres ou d'évaluation des dommages par les experts d'assurance. La proposition de loi retient plusieurs axes évoqués dans le rapport de la mission d'information : la réforme du fonctionnement du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds Barnier, le renforcement des droits des assurés et du montant des indemnisations dont ils bénéficient, la création d'un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques, le passage au niveau législatif de l'existence de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle, et enfin, la création, dans chaque département, d'une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle. On ne peut que souscrire à ces propositions dans leurs objectifs. L'article 1 prévoit de réformer le fonctionnement du fonds Barnier et, notamment, d'améliorer la stratégie de prévention des risques au sein dudit fonds. Les chiffres étayés par notre collègue Jean-François Husson insistent sur la nécessité d'augmenter les plafonds de ressources de ce fonds. Nous entendons cet argumentaire, qui s'inscrit dans une démarche pragmatique et de bon sens, tout comme nous pourrions aussi entendre celui qui incite au déplafonnement du fonds par souci de justice et d'efficacité. Cela étant, il me semble que c'est toute la doctrine du fonds Barnier que nous devrions revisiter au vu des enjeux climatiques auxquels nous De même, je crois que nous devons faire attention aux fausses bonnes idées quant à la composition du conseil de gestion. La prise de décision doit être efficace, sans se perdre dans des jeux d'intérêts complexes ; je soutiens à ce titre une instance de pilotage resserrée. Compte tenu des enjeux, nous devrions donner au conseil de gestion les moyens de son efficacité. Concernant l'article 2 relatif aux droits des assurés, je souligne, comme l'a fait la commission des finances, que le délai de prescription actuel de deux ans en cas de catastrophe naturelle encourage la mise en oeuvre rapide des travaux de réparation et qu'il ne pose à l'heure actuelle aucune difficulté pratique. Sur un autre point de l'article concernant l'intégration des frais de relogement d'urgence dans le périmètre de la garantie CatNat, il est vrai qu'il s'agit d'une demande forte des sinistrés, car la prise en charge du relogement est facultative et effectuée selon des modalités variables d'un assureur à l'autre.

Sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, je souscris aux dispositions de l'article 4 qui prévoient de rendre publics les rapports d'expertise utilisés par la commission interministérielle. Tout ce qui participe de la transparence de la décision publique représente en effet une avancée. avancée. Concernant les modalités de travail de cette commission, il faut éviter de rendre obligatoire sa consultation. Dans certaines situations, le caractère anormal du phénomène est malheureusement devenu évident.

Cette proposition de loi rappelle que, dans tous les cas, ce sont les maires qui sont en première ligne et qui fournissent la première réponse lorsqu'une catastrophe naturelle touche notre pays. Le texte, nous le savons, pourra être amélioré durant la navette parlementaire, certains points relevant par exemple du domaine réglementaire plutôt que de la loi. Nous sommes- pour beaucoup d'entre nous -malheureusement, et toujours en appui aux maires, confrontés dans nos territoires à ces situations qui nécessitent la mise en oeuvre du régime d'indemnisation. Je pense notamment à nos collègues des départements touchés régulièrement par les inondations. Cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte bien différent de celui de 1982, à une époque où les risques climatiques étaient sans doute moins nombreux aussi l'augmentation du nombre de phénomènes climatiques extrêmes et l'artificialisation des sols sont aujourd'hui responsables de bien des situations. Un quart des Français sont exposés à un risque d'inondation. La sécheresse ou ses conséquences touchent la quasi-totalité de notre territoire, et les risques de submersions marines ou d'érosion du trait de côte augmentent de façon considérable en métropole, mais aussi dans les territoires ultramarins.

C'est pourquoi des réponses pragmatiques doivent s'inscrire dans un ensemble de politiques publiques pour réaliser l'adaptation de notre pays aux évolutions climatiques. Il importe donc de prendre du temps et de poursuivre le travail en ce sens pour aboutir au dispositif le plus opérationnel possible. La parole est

Cette mission correspondait au domaine de compétence attribué à notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dont, d'ailleurs, le président et la rapporteure étaient membres. Nous étions 27 sénatrices et sénateurs issus de plusieurs commissions et de toutes sensibilités.

et l'autre dans le département de la Charente, où nous avons constaté le désarroi de nombreuses familles de sinistrés comme dans bon nombre de territoires français. La présence de nos collègues a été très importante, tant pendant les auditions que dans les déplacements. Cela prouve, madame la secrétaire d'État, que le sujet mérite de la part du Gouvernement une attention particulière, une écoute et la mise en oeuvre rapide des propositions qui sont issues de cet important travail, traduites dans la proposition de loi en discussion aujourd'hui. Nicole Bonnefoy propose ainsi un certain nombre de dispositifs améliorant le régime CatNat actuellement en vigueur. Madame la secrétaire d'État, les sujets des inondations et des vagues de submersion

nous attendons une réponse précise de la part de la ministre de la transition écologique et solidaire, Mme Borne, puisque nous avons, Nicole Bonnefoy et moi-même, cosigné un courrier lui demandant ce que le Gouvernement compte faire sur les mesures proposées dans le rapport de notre mission et qui relèvent du champ réglementaire, courrier resté pour l'instant sans réponse. En revanche, les catastrophes naturelles dues à la sécheresse sont particulièrement mal traitées et ont malheureusement conduit à de très nombreux drames humains dans plusieurs régions. Beaucoup de nos concitoyens dont les biens concernés n'ont pas été reconnus dans des périmètres de catastrophe naturelle les ont perdus ; c'est souvent le cas qui était, pour nombre d'entre eux, le fruit des économies de leur vie, madame la secrétaire d'État. Le Gouvernement ne peut pas laisser cette situation en l'état D'ailleurs, un ministre de votre gouvernement s'en est rendu compte, puisque M. Darmanin s'est permis de dégager des moyens financiers importants pour les sinistrés qui ont subi la sécheresse dans son département. Cela prouve des dysfonctionnements de l'État et des traitements inéquitables. L'inégalité de traitement de nos concitoyens, selon qu'ils ont ou non près de chez eux un ministre du budget est, vous en conviendrez, particulièrement anormale. Cette proposition de loi reprend des mesures proposées dans le rapport qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, a été voté à l'unanimité des groupes politiques du Sénat.

C'est la raison pour laquelle je vous appelle à soutenir le texte initial sur le déplafonnement du fonds Barnier et à ne pas voter l'amendement de plafonnement, puis à adopter les différents articles de cette proposition de loi tant attendue par les élus et par nos territoires.

Sachez également anticiper l'accélération du nombre et de la violence des catastrophes naturelles. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je crois profondément que c'est par la cohérence de nos travaux que nous pourrons petit à petit reconquérir la confiance de nos concitoyens. Les élus doivent faire preuve de courage et de ténacité face à une administration, notamment celle de Bercy, qui n'a souvent qu'une approche technocratique. J'en veux pour preuve le blocage des indemnisations des propriétaires du « Signal » malgré la loi Mes chers collègues, madame la secrétaire d'État, le courage est le prix de la dignité. Cela s'applique particulièrement au sujet d'aujourd'hui.

La seconde pensée, amicale, s'adresse à Nicole Bonnefoy et à mes collègues membres de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de nos régimes d'indemnisation, dont les travaux ont abouti Quand, dans le département de l'Aude, le temps est aujourd'hui péniblement à la reconstruction, notre proposition apporte des réponses concrètes aux problématiques rencontrées. Je concentrerai donc mon propos sur les articles 4 et 5 de ce texte. En plus de réformer la composition de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle, l'article 4 renforce les pouvoirs des maires. Vous l'aurez compris, apporter un soutien aux élus qui sont en première ligne lors de la survenance d'un tel événement est primordial. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du maire de déposer une demande de reconnaissance communale et d'informer les sinistrés de son avancement. De fait, les maires sont souvent mis en cause injustement face à la lenteur de l'instruction des dossiers, voire à la suite d'une décision de non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À cela s'ajoute une triste réalité : les élus, souvent livrés à eux-mêmes, ne bénéficient pas nécessairement d'informations précises ou de l'ingénierie leur permettant de gérer au mieux certaines situations. C'est donc une double peine à laquelle il nous faut impérativement nous attaquer en apportant un soutien et des outils aux élus dans la gestion de leurs dossiers CatNat. C'est pourquoi d'une part, allonge de dix-huit à vingt-quatre mois le délai pendant lequel une demande de reconnaissance peut être formulée après la survenance d'une catastrophe naturelle, les conséquences de certains événements climatiques n'étant pas nécessairement décelables immédiatement.

Délivrer une information complète aux maires, c'est ce qui a péché dans l'Aude. Notre rapport d'information a bien mis en avant l'esseulement des édiles lors de la survenance d'aléas climatiques exceptionnels. Cette situation est particulièrement difficile lorsqu'elle les expose directement à des sinistrés désemparés, voire lorsque les maires sont eux-mêmes sinistrés. Il leur revient pourtant de devoir expliquer l'état de la situation à leurs administrés et de se faire le relais de décisions ministérielles parfois difficile à entendre. L'article 5 entend remédier à cet isolement en instaurant dans chaque département une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle, laquelle permettra de les soutenir, de les accompagner dans leurs démarches, de les orienter devant un refus de reconnaissance et de les conseiller, le cas échéant. Enfin, il est un point sur lequel j'entends insister : la situation assurantielle des sinistrés. Dans l'Aude, certaines assurances refusent de reconduire des contrats souscrits avant la survenance d'une catastrophe naturelle, ou alors le font avec un malus exorbitant. C'est purement scandaleux. Il n'existe pas de moyens légaux pour les pour les contraindre, sinon le dispositif que propose l'article 4. Il supprime en effet la possibilité de moduler des franchises à la charge des assurés en fonction de l'existence d'un plan de prévention des risques naturels. Un dernier mot relatif au crédit d'impôt créé par l'article 3. Cette incitation est bienvenue, sinon indispensable. Néanmoins, comme son nom l'indique, le crédit d'impôt ne vaut que pour les gens qui payent des impôts. Que faire pour les autres ? Comment renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste pour les particuliers qui ne sont pas imposables sur le revenu ? La mécanique parlementaire est fortement contrainte et ne nous permet pas, madame la secrétaire d'État, de créer des subventions. Il est de votre responsabilité de les mettre en place. Nous comptons sur vous. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte apporte des réponses non exhaustives aux problématiques soulevées par les travaux de notre mission. Je vous invite à le voter unanimement. La parole

face aux aléas climatiques qui touchent nos territoires dans leur diversité, nous ne devons tolérer aucun fatalisme. Nous devons plutôt tirer les leçons des intempéries pour en finir avec les approches bureaucratiques dans la gestion des catastrophes naturelles. En effet, la pratique met en lumière des dispositifs sous-dimensionnés pour venir rapidement en aide aux sinistrés et aux collectivités. Comme le montrent les intempéries qui frappent régulièrement le sud-est de la France, et tout particulièrement le département des Alpes-Maritimes, l'aléa climatique est de plus en plus répétitif, violent et même meurtrier. La fin de l'année 2019 aura été particulièrement difficile pour un grand nombre de communes de mon département. S'agissant de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, s'il convient de saluer le travail des maires, qui se mobilisent pour enclencher la procédure auprès des services de l'État, la méthode de fonctionnement actuelle reste à géométrie variable. Son opacité fait naître de l'incompréhension, parfois même un sentiment d'injustice dans nos territoires. Je prendrai pour exemple les coups de mer d'octobre 2018 qui ont entraîné de fortes inondations dans les dans les Alpes-Maritimes. Les arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris pour certaines communes et pas pour d'autres, alors même que les dégâts étaient tout aussi importants. Lors de nos auditions dans le cadre de la mission d'information préfigurant cette proposition de loi, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre un avocat spécialisé

Les services des ministères pourraient ainsi se déplacer afin de décentraliser la décision interministérielle prise

parler de l'accompagnement des élus confrontés à la lenteur des procédures après une catastrophe. L'engagement et le courage des élus volontaires dans la gestion du risque doivent être valorisés par l'État, surtout lorsque leurs décisions permettent d'anticiper l'intervention de régimes d'assurance devenus obsolètes.

auteure de cette proposition de loi, qui a fait preuve d'un engagement particulièrement vigoureux, passionné et éclairé sur le sujet de la nécessaire réforme du régime des catastrophes naturelles. Permettez-moi, en propos liminaire, de témoigner, en tant que président du groupe interparlementaire d'amitié France-Australie au Sénat, de notre totale solidarité avec nos amis australiens, qui vivent un cauchemar absolu. Les chiffres sont terribles 10 millions d'hectares de végétation détruits, dont 800 000 hectares dans un seul incendie ; 2 000 maisons détruites ; 28 personnes y auraient trouvé la mort depuis septembre 1,25 milliard d'animaux auraient péri dans ces incendies. Le nuage provoqué va faire, selon les experts de la NASA, le tour de la planète. Tout cela résulte d'une sécheresse exceptionnelle sévissant depuis septembre sur l'île-continent. Hormis quelques invétérés et indécrottables climatosceptiques, chacun, et surtout les scientifiques, s'accorde pour nous alerter sur la croissance quasi exponentielle de l'intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles.

aux cyclones ou aux échouages massifs d'algues sargasses sur les littoraux antillais, en passant par des phénomènes fréquents de sécheresse dans nombre de nos départements, notre pays, la France,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pas un pays dans le monde n'est épargné par une augmentation significative des catastrophes naturelles, dans leur fréquence et dans leur intensité. L'Australie en proie aux flammes, les dernières inondations en Indonésie : il n'est plus possible de nier l'évidence du dérèglement climatique et de ses conséquences. La France, notre pays, connaît régulièrement son lot de catastrophes naturelles. Je pense aux récentes inondations meurtrières qui ont touché le sud de la France, mais également aux tempêtes qui ont frappé nos côtes métropolitaines et nos outre-mer. Aujourd'hui encore, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique ont été placés en vigilance orange pour risque de « vagues-submersion » et « pluie-inondation Ces phénomènes, nous devons désormais apprendre à vivre avec et à les anticiper : cela s'appelle la résilience. C'est en Vendéen qui a connu la tempête Xynthia que je vous le dis. Je salue de nouveau le travail de nos collègues, Nicole Bonnefoy, auteure de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, et Michel Vaspart, dans le cadre de la mission d'information, dont le rapport a été adopté à l'unanimité. Comme je l'avais souligné lors du débat consacré à ce sujet, voilà peu, dans cet hémicycle, nous devons adopter une réelle culture du risque qui permette à notre pays de mieux appréhender ces événements. Bien entendu, je ne peux qu'être en accord avec l'idée de déplafonner le fonds Barnier. Depuis sa création, le champ d'action de ce fonds n'a cessé de s'élargir, mais ses moyens d'action n'ont pas cessé, quant à eux, de diminuer. le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, a été prélevé de 55 millions d'euros en 2016 et de 70 millions d'euros en 2017. Lors de l'examen de la loi de finances pour 2018, le Gouvernement a également décidé de plafonner ce fonds à hauteur de 137 millions d'euros, alors que les recettes, issues des cotisations des assurés, sont supérieures à 200 millions J'étais intervenu dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 pour rétablir les moyens du fonds Barnier. Malgré un vote quasi unanime d'un amendement déplafonnant le fonds, le Gouvernement n'avait pas souhaité le conserver dans le texte définitif. L'an dernier, le projet de loi de finances pour 2019 est de nouveau venu diminuer de 20 millions d'euros le montant des dépenses autorisées pouvant être consacrées au financement des études et des travaux de prévention par les collectivités territoriales. Là encore, nous avions dénoncé cette ponction L'automne dernier, nous avons déposé sans succès, avec Michel Vaspart, des amendements, déclarés irrecevables, demandant de nouveau le déplafonnement du fonds. Il y a donc un réel paradoxe entre cette nécessité de préparer la France à ces changements climatiques et les faibles moyens, de surcroît en diminution, qui y sont consacrés. C'est donc en toute logique que je soutiens le déplafonnement, dont nous allons débattre dans quelques instants. L'argent des assurés, destiné à financer le fonds de prévention, doit être pleinement utilisé pour cet objet. Je soutiens également l'idée d'un élargissement des affectations de ce fonds, qui est aujourd'hui un levier sous-utilisé dans le secteur de la prévention. Au-delà de cette proposition de loi, j'appelle le Gouvernement à définir, avec les acteurs concernés, une véritable stratégie nationale de prévention des risques naturels, comme il en existe déjà dans de nombreux pays. Madame la secrétaire vous avez évoqué à deux reprises dans votre intervention le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, dont c'est la vocation de travailler avec les différents acteurs, d'analyser les phénomènes et de définir la stratégie. Je vous invite à le réunir rapidement, très rapidement, j'y insiste, car il ne s'est,

seront intégrées à notre concertation. Il y a les éléments qui sont législatifs, sur lesquels nous travaillons, et les éléments réglementaires, qui viendront en complément, évidemment en miroir, pour que l'ensemble soit cohérent. Madame Sollogoub, l'extension des délais dont bénéficient les assurés pour déposer leur demande d'indemnisation fait partie des mesures que nous voulons soumettre Je ne peux pas encore vous dire si c'est vingt jours, trente jours, mais, en tout état de cause, on voit bien que le délai de vingt jours est un minimum. Nous sommes également très favorables à une meilleure prise en compte du risque sécheresse dans les zones de construction. C'est ce que permettent les textes d'application de la loi ÉLAN. Pour répondre à je vous indique que le décret du 22 mai 2019 rend obligatoire l'étude de sol à compter du 1 janvier 2020 pour la construction de maisons individuelles sur des terrains exposés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles dans les zones à exposition moyenne ou forte. Voilà pour les quelques précisions à apporter. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Dans ces conditions, je me verrai dans l'obligation de lever la séance une fois ce délai épuisé. Si nous n'avons pas achevé l'examen du second texte, il appartiendra à la conférence des présidents d'inscrire la suite de la discussion de cette proposition de loi à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Bonhomme, sur l'article. Cette proposition de loi de Nicole Bonnefoy reprend un certain nombre de propositions du rapport de la mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution des régimes d'indemnisation. À cet égard, les maires, en particulier, savent combien la recrudescence et l'intensification des phénomènes de catastrophes naturelles est un enjeu majeur pour un nombre de plus en plus important de nos concitoyens. En effet, ils ont eu à en gérer les conséquences pour des sinistrés qui se trouvent parfois dans des situations absolument dramatiques. C'est pourquoi il est essentiel d'apporter une réponse rapide et concrète, avec un renforcement de l'indemnisation, mais également d'améliorer la prévention, notamment à travers une incitation fiscale pour la réalisation de travaux. L'article 1 de la proposition de loi comporte plusieurs dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs, plus communément appelé fonds Barnier. On peut, à bon droit, opter pour le déplafonnement du montant des recettes affectées au fonds, puisqu'il est principalement financé par un prélèvement obligatoire de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles payées par les assurés au titre de la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. À tout le moins, l'augmentation des recettes du fonds me paraît nécessaire.

nombre de propos qui viennent d'être tenus au cours de la discussion générale. Bien sûr, je voudrais reprendre à mon compte l'intervention de mon collègue François Bonhomme sur le déplafonnement du fonds Barnier. On a eu l'occasion d'en discuter. J'ajoute deux réflexions qui me paraissent essentielles. Je viens d'un département qui a vécu, voilà un peu plus de deux mois, un séisme d'une ampleur assez inédite sur le territoire hexagonal. Les maires, notamment, sont en première ligne pour gérer les conséquences de

qui sont prélevées sur les assurances, et elles devraient être utilisées en totalité. Il n'empêche que des gouvernements, de majorités différentes, ont

de fixer le plafond à 200 millions d'euros pour l'année 2020, ce qui, on le sait, répondra aux besoins.

doit nous conduire à travailler, sous l'autorité du Gouvernement, à l'amélioration du fonctionnement de tous ces dispositifs. C'est la raison pour laquelle

Nous partageons l'idée qu'il importe de donner des moyens suffisants en soutien des mesures de prévention et de traitement des vulnérabilités, notamment via le fonds Barnier.

Nous prenons acte de vos propositions, que nous allons étudier, sachant que toute évolution budgétaire du fonds a vocation, de notre point de vue, à être discutée en loi de finances. Cet aspect méthodologique me conduit à donner un avis défavorable

présenter l'amendement n° 6. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, deux amendements identiques ont été adoptés par le Sénat sur l'initiative de nos collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart, afin de supprimer plusieurs sous-plafonds de dépenses du fonds de prévention des risques naturels majeurs, et de donner davantage de souplesse dans la gestion de ce fonds.

L'article 81 de la loi de finances pour 2020 a supprimé plusieurs sous-plafonds de dépenses du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Dans la même logique, cet amendement vise à supprimer le sous-plafond de 5 millions d'euros applicable au financement des frais de démolition des locaux à usage d'habitation informels, exposés à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dans les départements et régions d'outre-mer, et des aides financières versées aux occupants de ces habitations, la possibilité de financer ce type de dépenses par le fonds ayant été étendue jusqu'en 2024 par l'article 232 de la loi de finances pour 2020.

avoir pour effet de réduire la vulnérabilité de leurs biens à usage d'habitation ou de leurs biens professionnels aux risques naturels majeurs.

pour réclamer à leur assurance le règlement de l'indemnisation qui leur est due en cas de dommages résultant de catastrophes naturelles. Si cette prescription biennale est suffisante pour des dommages immédiats résultant d'aléas naturels comme les inondations, les séismes ou les avalanches, qui nécessitent des réparations urgentes, tel n'est pas forcément le cas des dommages résultant des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, qui peuvent apparaître dans un temps plus long. Le présent amendement tend à limiter l'allongement du délai de prescription de deux à cinq ans aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

aux assurés doivent permettre « un arrêt des désordres existants [ ...], en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles ». Il s'agit de faire en sorte que les réparations réalisées à la suite d'un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse tiennent compte des meilleures techniques disponibles, afin qu'elles soient le plus durables possible.

Toutefois, ces amendements n'ont pas de valeur ajoutée par rapport au droit en vigueur : le mécanisme assurantiel en matière de catastrophes naturelles, comme pour l'ensemble des contrats d'assurance, est fondé sur le principe indemnitaire fixé à l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel la réparation doit être proportionnelle au préjudice causé. Les travaux de réparation sont réalisés selon les normes en vigueur, en particulier en matière de construction. Au passage, je me réjouis de l'adoption de l'ensemble des textes d'application de la loi ÉLAN, qui permettront de renforcer la résilience du futur bâti. Il n'est pas envisageable que les assureurs indemnisent au-delà du préjudice subi, notamment en vue de prévenir de futurs sinistres, car cela ne relève pas de leur responsabilité.

n° 12 rectifié. Cet amendement concerne les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées. Il vise à préciser que cette prise en charge pourra être sollicitée lorsque le bien endommagé constitue la résidence principale du sinistré, et que celle-ci est insalubre ou présente un danger pour la sécurité de ses occupants. Cette précision est importante.

En tout état de cause, si une prise en charge est retenue, il sera nécessaire d'encadrer ses modalités, notamment de la limiter aux sinistrés qui en ont réellement besoin, conformément à l'esprit de cet amendement- le fait que le bien Nous engagerons une concertation spécifique sur ce point, afin d'affiner le dispositif et, notamment, les conditions dans lesquelles cette prise en charge pourra être effectuée dans un cadre budgétaire maîtrisé. Pour

des risques naturels, la réduction d'impôt apportée à hauteur de 18 %, voire de 26 %, des travaux de confortement contre les risques sismiques ou cycloniques réalisés par les particuliers sur les logements anciens affectés à la résidence principale et qui sont situés outre-mer. Même avec les précisions apportées par votre amendement, le texte ne définit pas suffisamment les modalités d'application de ce crédit d'impôt pour être considérée comme fixant des règles d'assiette de l'impôt au sens de l'article 34 de la Constitution. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

il vise à supprimer la mention selon laquelle l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut être pris que sur la base des travaux de la commission interministérielle CatNat. Je précise cela par rapport aux remarques formulées plus tôt. Il convient en effet de laisser la possibilité au Gouvernement, en cas d'urgence, de constater l'état de catastrophe naturelle sans que la commission interministérielle se soit réunie au préalable.

de cette algue. Vous pouvez aller naviguer sur tous les sites internet et voir à quoi cela ressemble. La mer devient complètement impénétrable, les plages également. Nous vivons,

naturelles, chargée de donner un avis consultatif sur chaque dossier communal transmis par les préfets de département. C'est sur le fondement de ces avis que les ministres compétents décident de la reconnaissance ou non des communes en état de catastrophe naturelle. Son rôle est donc singulier et revêt une importance particulière pour le sort de nos territoires. Il serait opportun que cette commission intègre des représentants du ministère de la transition écologique et solidaire. En effet, avec le réchauffement climatique, nous assistons déjà à la multiplication de phénomènes naturels et météorologiques extrêmes. Il serait utile que le ministère de la transition écologique puisse participer aux travaux de cette commission.

à certaines conditions : la commission doit demeurer une enceinte consultative, technique, et ne doit rendre que des avis simples. Cependant, le Gouvernement partage le souhait d'une transparence de la commission interministérielle relative aux catastrophes naturelles afin de ne laisser aucun doute aux sinistrés sur l'objectivité des avis proposés. Il est notamment envisagé de refondre les circulaires et instructions existantes encadrant la procédure en une seule circulaire interministérielle détaillant les modalités de mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Publiée au, impérative, opposable et contrôlée par le juge administratif, cette circulaire pourrait préciser la composition exhaustive de la commission et son fonctionnement. S'agissant du sous-amendement n° 26 rectifié, le Gouvernement comprend et partage la préoccupation des sénateurs concernant le phénomène des algues sargasses. Toutefois, ce sous-amendement ne nous semble pas constituer une réponse appropriée. Il remet en cause le fondement même du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. La définition d'une catastrophe naturelle est encadrée depuis la création de ce régime. C'est le caractère anormal du phénomène qui constitue la base de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Revenir sur cette définition déstabiliserait l'ensemble de ce système qui a prouvé maintes fois sa légitimité. En l'état actuel de sa rédaction, le code des assurances n'empêche pas la reconnaissance en état de catastrophes naturelles des communes sinistrées par un phénomène inédit, dès lors qu'il présente un caractère anormal. un caractère anormal. La cause directe des dommages causés par les algues sargasses n'est pas le phénomène d'échouage lui-même, mais c'est la décomposition de ces dernières du fait de leur non-enlèvement des plages. C'est l'absence de relation directe entre le phénomène et les dégâts recensés qui explique le rejet des demandes communales de reconnaissance. Par ailleurs, même si le Gouvernement décidait de reconnaître en état de catastrophes naturelles les communes touchées par l'échouage massif d'algues marines, cette reconnaissance serait sans effet sur la situation des collectivités, des particuliers et des entreprises. Les collectivités locales n'étant pas assurées pour les biens éventuellement endommagés par l'échouage des algues, elles ne seraient pas indemnisées à ce titre. S'agissant des particuliers et des entreprises, seuls seuls les dommages aux biens sont pris en charge par les assureurs dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles. S'agissant des entreprises, certains biens sont exclus du régime des catastrophes naturelles dans la mesure où ils relèvent d'autres régimes spécifiques d'assurance. Or ce sont peut-être ces biens-là qui sont touchés par les sargasses. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable

madame la ministre,

est ainsi libellé : La parole est à Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à préciser que, en cas de refus de leur première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les communes disposent d'un délai de six mois pour présenter une nouvelle demande assortie d'éléments techniques complémentaires. C'est très important pour les communes, en particulier pour les petites communes. Gouvernement ? Le réexamen des demandes de reconnaissance rejetées par arrêté existe déjà. Dans le cadre de recours gracieux, des expertises complémentaires peuvent être sollicitées par le ministère de l'intérieur auprès des organismes d'expertise de l'État compétents.

Cette proposition tend à modifier l'objet des cellules de soutien qui visent aujourd'hui à partager l'expérience entre élus locaux et personnalités qualifiées. Cette rédaction est susceptible d'introduire de la confusion avec les missions du préfet du département et les services de l'État dans le suivi post-crise à l'échelle départementale. Sur le fond, l'idée de cellules de soutien semble intéressante. Son organisation pratique pose cependant la question de son articulation avec les services de l'État et du préfet du département. J'émets donc un avis défavorable, mais je suis d'accord pour travailler sur le sujet. Je mets aux voix l'amendement

je tiens avant tout à remercier notre rapporteure, Nadine Grelet-Certenais, de la grande qualité de son travail sur la présente proposition de loi dont elle est co-autrice. « Uber est le symbole d'un changement social irréversible » déclarait en 2015 son directeur général. C'est en tout cas ce que cette plateforme numérique et ses pareilles veulent nous faire croire. Ce faisant, elles prétendent nous imposer un nouveau contrat social avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Ce contrat présuppose notamment que le droit du travail soit soumis aux impératifs d'un certain type de modèle économique être contourné par tout moyen possible, y compris par le biais du subterfuge numérique. Pour notre part, au groupe socialiste et républicain, nous rappelons que notre organisation sociale repose sur un dogme juridique, porteur de valeurs. Ces valeurs, dont nous avons fait le choix, avec le Conseil national de la Résistance, ont présidé à la formalisation de notre ordre social et économique. L'article 1 de notre Constitution dispose ainsi : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Elle est donc sociale ! Il n'y a pas de fatalité à subir les failles de notre système ni les choix d'acteurs ultralibéraux quand ils minent ce modèle et en remettent en cause les fondamentaux. Ces fondamentaux sont pourtant mis à mal par un type d'intermédiation qui a émergé avec l'économie 2.0. L'intervention d'un tiers dans la relation salariale traditionnelle, qui unit de manière directe le salarié et son employeur, a été longtemps interdite en France. Il s'agissait d'empêcher les pratiques de marchandage ou les prêts de main-d'oeuvre lucratifs par lesquels des intermédiaires s'immisçaient pour « revendre » le travail des ouvriers. Ce n'est qu'à partir de 1972 que cet interdit a été levé. L'intermédiation s'est en effet révélée prometteuse pour répondre aux défis de l'emploi. S'il ne s'agit pas encore d'un phénomène massif dans notre pays, l'utilité des acteurs de l'intermédiation est démontrée. Celle-ci permet, par exemple, la mise en place de nouvelles formes de protection de travailleurs victimes de précarité dans le cadre de leur expérience professionnelle ; les coopératives d'activité et d'emploi (CAE) en font partie. cette logique est dévoyée par des entreprises qui ont conçu un modèle de plateformes numériques exposant les travailleurs à la précarité. Ces entreprises font le choix d'organiser leur modèle économique autour de l'utilisation d'algorithmes, qui rebattent les cartes du secteur de l'intermédiation. Elles se sont structurées de façon à tirer profit des failles d'un système de protection sociale qui se veut protecteur des travailleurs. Le recours abusif aux auto-entrepreneurs et l'utilisation d'algorithmes sont les moyens favorisant l'exploitation de ces failles. ces organisations du versement de cotisations sociales, alors même que leur modèle économique est si peu viable que le paiement de salaires en bonne et due forme les mènerait à la banqueroute Le récit de la révolution numérique et des nouveaux mondes que celle-ci ouvrirait vient achever l'opération de camouflage d'une entreprise prosaïquement opportuniste et niant les droits des travailleurs. Ce subterfuge numérique, c'est l'invocation incantatoire des intelligences artificielles, qui remplaceraient le travailleur humain. derrière ces intelligences artificielles, ce sont des individus qui travaillent, trop souvent dans la précarité et pour des missions mal payées. Ce subterfuge, c'est aussi le recours, par les plateformes dominantes, à la poudre aux yeux des algorithmes.

opacité. Ils génèrent des conditions de travail instables et une rémunération volatile, sources de souffrance au travail. Si l'activité des plateformes qui y recourent s'inscrivait dans l'esprit de notre République sociale, ces conditions seraient établies dans des contrats à même d'offrir de la prévisibilité aux travailleurs. Or tel n'est pas le cas les travailleurs concernés sont exposés à une relation commerciale structurellement inégalitaire. Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs sont dépouillés de leur droit à négocier les conditions dans lesquelles ils effectuent leurs prestations ainsi que leurs rémunérations. Je parle des professionnels qui ont voulu faire le choix de l'autonomie, Une partie d'entre eux ne veut pas revenir dans le cadre protecteur du salariat, jugé trop contraignant. Ces travailleurs se trouvent pourtant aujourd'hui, contre leur gré, dans une situation de dépendance et de subordination de fait, situation qui, justement, définit la condition salariale. Dépouillés de leurs droits sociaux, ils n'ont cependant ni les avantages ni la protection de l'indépendance. Ils sont pourtant combatifs ; ils ont su, malgré leurs contraintes professionnelles, faire émerger une problématique jusque-là méconnue. Nous les remercions pour leur rôle de lanceurs d'alerte ils donnent à la société l'occasion de se saisir d'une situation d'injustice et de mettre fin à des pratiques entrepreneuriales qui représentent un danger pour notre société. Je pense aux chauffeurs de VTC, qui peuvent être victimes de déconnexions abusives

Ces plateformes ne font donc rien de moins que de remettre au goût du jour le tâcheronnage, en le revêtant des habits scintillants du progrès technique et des mirages numériques. Pour l'instant, le capitalisme de plateformes n'a pas permis de servir l'intérêt général. Le travail que nous avons mené sur le sujet nous a au contraire conduits à la conclusion opposée. Peu de sphères de notre société pourraient se targuer d'être à l'abri des bouleversements induits par ce nouveau type d'organisation économique. De très nombreux secteurs de notre économie de service sont susceptibles d'être « ubérisés », selon le terme désormais consacré. Il n'est pas un secteur qui ne soit susceptible de faire l'objet de cette révolution délétère. Face à ce constat, nous avons tiré des conclusions. Nous considérons que la société ne doit pas fermer les yeux sur le détournement de son système de protection sociale à des fins privées, mettre à bas les droits des travailleurs, ni piller les caisses de la sécurité sociale pour garantir à des entreprises une viabilité qui n'est nullement acquise. Certes, en France, comme à travers le monde, la justice a été saisie à plusieurs reprises pour mettre fin à des situations d'abus caractérisé. Ainsi, Deliveroo est en butte en France à des actions de ses livreurs, qui contestent un changement de tarification opéré en juillet.

À la suite de cet arrêt, tous les chauffeurs ou livreurs auto-entrepreneurs se sont trouvés en mesure de demander une requalification de leur contrat commercial en CDI, la requalification des salariés déguisés en salariés de plein droit étant rétroactive. Les plateformes se sont trouvées confrontées au risque de devoir verser des cotisations sociales qu'elles n'avaient sans doute pas provisionnées. Les conséquences financières de cette décision sont potentiellement énormes, notamment au profit de l'Urssaf. L'une des réactions des plateformes à ces décisions consiste en la mise en place de mesures qui ne valent que par leur effet d'annonce. Deliveroo a ainsi annoncé, en octobre 2019, la mise en place, pour ses livreurs, en France, d'une assurance maladie complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il s'agit, selon les principaux intéressés, d'un simple effet d'annonce ... Les recours juridictionnels et le droit existant nous paraissent donc insuffisants pour faire face à la nature et à l'ampleur des bouleversements qu'est susceptible d'induire l'économie de plateforme, d'autant que nous sommes confrontés à une démarche gouvernementale visant à exempter les entreprises de leurs devoirs en tant qu'employeurs. Je fais ici référence à l'inscription par le Gouvernement de chartes facultatives dans la loi Mobilités, qui disposait, dans son article 20, que les plateformes de livraison peuvent instaurer de telles chartes, qui seraient porteuses de droits sociaux. Cette parade vise à soustraire les plateformes à d'éventuelles requalifications des contrats des travailleurs indépendants en salariat.

nous proposons une réponse législative dédiée à cette problématique, mais il n'est pas question d'infléchir le droit du travail pour donner à des entreprises au modèle économique non rentable accès à des travailleurs bénéficiaires de droits au rabais et, donc, moins coûteux.

Il s'agit de réaffirmer des valeurs profondément progressistes de défense du droit du travail et de la citoyenneté sociale des travailleurs. C'est aussi pour nous l'occasion de mettre en valeur le modèle coopératif, qui repose sur la propriété collective d'un outil de production et sur la participation démocratique des coopérateurs aux décisions de l'organisation. Ce modèle résout le problème de l'indépendance, revendiquée par les travailleurs par les travailleurs numériques ou, en tout cas, par leurs « représentants ». L'entrepreneur salarié dispose des mêmes protections sociales qu'un salarié et d'un accompagnement de la coopérative pour la gestion administrative. En ce qui concerne son salaire, il reçoit une rémunération composée d'une part fixe versée mensuellement et d'une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement liées à celle-ci et de sa contribution relative aux services mutualisés proposés par la coopérative. La présente proposition de loi constitue par conséquent une réponse législative sans ambiguïté face à la tentative des plateformes de contourner notre droit social conquis de haute lutte. Elle s'inscrit en défense du modèle social français.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Monique Lubin, que j'ai cosignée avec les membres du groupe socialiste et républicain, vise à rétablir les droits sociaux dont un nombre croissant de travailleurs sont privés, du fait du développement de l'économie des plateformes. En effet, si le numérique est porteur de nombreuses opportunités, il peut aussi représenter, pour notre cohésion sociale, une menace contre laquelle il est indispensable que les pouvoirs publics interviennent. Les différents travaux lancés au Sénat sur le sujet témoignent de la prise de conscience de cette nécessité. Si la commission des affaires sociales n'a pas adopté de texte, elle a reconnu l'importance de cette question et elle a partagé certains constats. L'apparition et le développement d'entreprises proposant de mettre en relation des travailleurs indépendants et des consommateurs des applications numériques représentent l'une des évolutions majeures du marché du travail depuis les années 2010. Si chacun a en tête les voitures de transport avec chauffeur et la livraison de repas, ce phénomène touche un nombre sans cesse croissant de secteurs : métiers du numérique, services à la personne, hôtellerie-restauration et jusqu'aux micro-tâches extrêmement parcellisées confiées à des « travailleurs du clic L'économie des plateformes concerne potentiellement un périmètre très large. Les informations sur la taille de cette économie restent toutefois, à ce jour, très incomplètes. L'estimation la plus répandue fait état d'environ 200 000 travailleurs actifs, à plein temps ou de manière plus ponctuelle. Il n'en reste pas moins que ce phénomène, de plus en plus visible, est révélateur d'une tendance inquiétante, dont la comptabilisation paraît constituer un enjeu en soi. Le développement des plateformes numériques de mise en relation vient à rebours d'une longue dynamique créatrice de droits. En effet, le mode de fonctionnement de ces plateformes consiste, en s'abritant derrière une indépendance parfois purement formelle, à s'affranchir des obligations que le code du travail impose aux employeurs vis-à-vis de leurs salariés, tout en éludant largement la participation au financement de notre système de protection sociale. Elles s'appuient pour cela sur les avantages fiscaux et sociaux et sur la simplicité du régime de la micro-entreprise, ainsi détourné de sa finalité initiale. Pour les travailleurs, l'illusion d'une autonomie et d'une liberté, ainsi que la préférence à court terme pour une rémunération plus élevée, se traduit en fait par une protection faible, voire inexistante, contre les risques d'accident du travail et de perte d'emploi, et par une absence de droits face au réel donneur d'ordres, notamment en matière de durée du travail. Ainsi, on peut voir dans le développement de l'économie numérique l'émergence d'une nouvelle forme de tâcheronnage. Ce phénomène ne doit pas être considéré isolément. Il s'agit du dernier avatar de la flexibilisation des rapports de travail, qui accentue la polarisation du marché du travail et ouvre la voie à une « hyper-précarisation » de certaines populations. Face à cette situation, le législateur a, jusqu'à présent, cherché à conférer aux travailleurs des plateformes des embryons de droits, dont une grande partie repose sur le bon vouloir des plateformes. Avec l'entrée en vigueur de la loi d'orientation des mobilités, les plateformes de VTC et de livraison ont désormais la possibilité d'établir unilatéralement une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale. Le Conseil constitutionnel, en censurant une partie de ces dispositions dans sa décision du 20 décembre dernier, a estimé que le législateur était allé trop loin dans l'abandon aux plateformes de l'exercice de sa compétence. Cette démarche témoigne à mon sens d'une timidité des pouvoirs publics à l'égard des opérateurs de plateforme qui n'a pas lieu d'être, s'agissant de défendre une certaine conception de notre modèle social. En outre, cette ébauche de cadre est source d'insécurité juridique, comme le prouve la jurisprudence récente de la Cour de cassation- le fameux arrêt du 29 novembre 2018 -établissant que les conditions dans lesquelles certaines plateformes se comportent à l'égard de leurs « partenaires » permettent d'établir l'existence d'un lien de subordination. D'autres pays ont eu plus de courage ; je pense à la loi adoptée en septembre dernier par l'État de Californie, berceau des plateformes, qui soumet au respect de conditions rigoureuses l'emploi de travailleurs indépendants. Cette proposition de loi adopte donc une démarche toute différente : son article unique remplace l'ensemble des dispositions de la septième partie du code du travail applicables aux travailleurs des plateformes par une règle simple, qui renvoie à des statuts préexistants et protecteurs au lieu de laisser prospérer un « tiers statut » incomplet. Il s'agit d'imposer aux plateformes d'avoir recours soit à des salariés directement, soit à des entrepreneurs salariés adhérant à une coopérative d'activité et d'emploi. Ces CAE sont apparues dans les années 1990 et ont été consacrées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'une forme originale de coopérative qui permet de concilier entrepreneuriat individuel et protection sociale. En effet, cette loi, dite « Hamon », a introduit dans la septième partie du code du travail un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée : le contrat d'entrepreneur salarié et associé. Le titulaire de ce contrat a un statut hybride susceptible de répondre aux besoins d'autonomie et de protection des travailleurs de plateformes : vis-à-vis des clients, l'entrepreneur salarié est un entrepreneur indépendant ; vis-à-vis de la coopérative, il est un salarié à part entière. Au-delà d'un statut, la CAE apporte au travailleur, en échange d'une contribution financière, un accompagnement dans son projet, des services mutualisés ainsi qu'un cadre collectif. Si elles restent méconnues, les CAE sont en plein développement. Certaines régions ainsi que des départements ont été des soutiens importants de leur constitution. Cette proposition de loi s'inscrit dans la lignée d'expériences conduites en France et en Europe qui visent à promouvoir un modèle alternatif en s'appuyant sur un fonctionnement coopératif. D'une part, à côté des plateformes de type capitalistique, d'autres types de plateformes émergent, parfois regroupées sous l'intitulé de « coopérativisme de plateforme Elles sont encore peu nombreuses en France, mais elles peuvent réussir, en se positionnant sur des niches que n'occupent pas, pour le moment, les grandes plateformes. D'autre part, l'idée de l'entreprise porteuse coopérative proposant aux travailleurs opérant sur les plateformes un statut de salarié tout en les laissant autonomes dans l'organisation de leur profession a directement inspiré la présente proposition de loi. Il existe à ce jour un précédent en Europe : l'expérience menée par la coopérative Smart, en Belgique, entre 2013 et 2017, auprès de coursiers à vélo. Cette expérience a permis de montrer qu'un tel modèle, très proche de celui de la CAE, pouvait aboutir à des résultats, en donnant à des travailleurs organisés sous forme de coopérative un pouvoir de négociation face aux plateformes. Elle a par ailleurs fourni de précieuses informations sur l'accidentologie des coursiers à deux-roues, confirmant le caractère particulièrement exposé de cette activité. L'objet de cette proposition de loi est donc non pas de sécuriser économiquement et juridiquement le modèle délétère promu par les plateformes, mais bien de promouvoir un modèle susceptible de répondre à la recherche d'autonomie des travailleurs, tout en offrant à ceux-ci un soutien juridique, une inscription dans un collectif et une protection sociale appropriée. Néanmoins, la commission des affaires sociales a considéré que les problématiques soulevées par le développement de l'économie des plateformes ne pouvaient trouver de réponse unique, en raison notamment de la diversité des acteurs et des situations, et que le salariat ne correspondait pas nécessairement aux aspirations de ces travailleurs. Elle n'a donc pas adopté la proposition de loi. Vous comprendrez que, à titre personnel, je le regrette ; tous les travailleurs devraient bénéficier d'une protection sociale digne de ce nom, y compris ceux qui ne le demandent pas. La commission a confié en septembre dernier à Michel Forissier, Catherine Fournier et Frédérique Puissat une mission d'information, qui doit rendre ses conclusions au printemps. Cette mission se poursuivra donc, enrichie des réflexions et des débats menés dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, étant entendu que nous visons tous le même but : la protection des travailleurs.

l'essor de l'économie des plateformes numériques de mise en relation de travailleurs avec les consommateurs est l'une des évolutions les plus importantes du marché du travail depuis une dizaine d'années, en France, en Europe et dans le monde.

très diverses. Notre conviction est qu'il n'y a pas de solution unique pour répondre à tous les défis de la construction d'une économie des plateformes financièrement soutenable, techniquement innovante et socialement responsable, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doive pas être socialement responsable. Or que prévoit votre proposition de loi ? D'abord, d'un point de vue légistique, elle supprime l'ensemble des dispositions du titre IV du livre III du code du travail ; il s'agit de la partie dédiée aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Je rappelle que cette partie du code du travail a été créée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et qu'elle a été complétée, très récemment, par la loi d'orientation des mobilités.

Votre proposition de loi, cela a été souligné lors de l'examen en commission, présente une double difficulté. En premier lieu, en créant une obligation générale, elle ne prend en compte ni la diversité des aspirations des travailleurs qui recourent aux plateformes ni la spécificité du projet porté par les coopératives d'activité et d'emploi. En effet, le champ des travailleurs des plateformes, tel que défini dans la proposition de loi, est très large, puisqu'il comprend tous les types de plateformes numériques, indépendamment de leur degré d'intervention dans les conditions d'exercice de l'activité. Or les utilisateurs des plateformes ne sont pas tous des travailleurs précaires ou des auto-entrepreneurs qu'il faudrait accompagner dans le lancement de leur activité. Certains sont des travailleurs en « »- pour le dire en bon français -très qualifiés ou des travailleurs indépendants bien installés, qui recourent aux plateformes pour trouver des clients ; adhérer à un projet coopératif ne répond pas forcément à leurs aspirations. Leur couverture sociale, qui pourrait, certes, être améliorée, correspond à celles des autres travailleurs indépendants et pose, plus largement, la question de la convergence de nos systèmes de protection sociale, ce que nous sommes en train de faire à propos des retraites. À l'autre bout du spectre, certains travailleurs ne recourent aux plateformes que de manière occasionnelle, comme revenu d'appoint ; ce sont des étudiants ou des salariés qui recherchent un complément de revenu. De la même manière, ce ne sont pas des entrepreneurs qu'il convient d'accompagner dans le lancement d'une activité, ce qui est l'objet même des CAE auquel vous proposez de recourir systématiquement. En second lieu, faire des coopératives un simple outil d'accès à la protection sociale le statut de salarié revient à en détourner l'objet.

ne fonctionnent que grâce à un fort dynamisme entrepreneurial et territorial, et elles impliquent l'adhésion des membres au projet porté. Le principe de l'obligation va à l'encontre de cet esprit d'adhésion. Cela dit, il y a d'autres voies possibles pour améliorer la protection sociale de ces travailleurs indépendants. Depuis 2016, le législateur s'est efforcé de construire la responsabilité sociale des plateformes. Des progrès importants ont été acquis pour ces travailleurs, en matière d'accident du travail, travail, de formation ou de droit d'action collective. Ainsi, la loi d'orientation des mobilités ainsi que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont notamment défini des règles d'alimentation du compte personnel de formation. Je rappelle par ailleurs que la loi sur les mobilités a mis en place le droit à la déconnexion et la transparence du prix des courses, pour les plateformes électroniques de mise en relation avec des VTC ou des coursiers. Quant aux chartes, homologuées par l'administration, elles ont vocation à inciter les plateformes à être plus transparentes sur leurs engagements sociaux et à leur laisser la possibilité d'aller plus loin. Enfin, sur le volet du dialogue social, des débats parlementaires avaient en effet fait émerger la nécessité d'organiser une meilleure représentation de ces travailleurs, afin de garantir à ceux-ci l'existence d'un dialogue équilibré avec les plateformes numériques, et de leur permettre ainsi de contribuer à la détermination de leurs conditions de travail. C'est précisément l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités. D'ailleurs, dans la perspective de l'élaboration de cette ordonnance, le Gouvernement a confié, hier, une mission à M. Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui sera accompagné d'experts pour travailler sur ce sujet. De façon générale, les travailleurs des plateformes posent la question de l'amélioration de la protection sociale des indépendants et celle de l'universalité de notre système de protection sociale. Plusieurs pas ont été faits ; j'en citerai deux depuis janvier 2019, les travailleuses indépendantes, chefs d'entreprise et conjointes collaboratrices bénéficient des mêmes prestations de maternité que les salariées et, depuis le 1 novembre 2019, les travailleurs indépendants ont droit à l'assurance chômage, sans cotisation supplémentaire. donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à rejeter cette proposition de loi, mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous retrouver prochainement sur le sujet du droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants, puisqu'il fait l'objet depuis septembre dernier de la mission d'information,

En réalité, nous avons bien affaire à des plateformes de travail. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs, depuis lors, confirmé cette analyse : la mise en relation n'est que l'accessoire de l'activité principale de ce type de plateformes, qui ne peuvent prétendre se présenter comme de simples plateformes de mise en relation.

? Nous pensons donc que, en l'état, ce texte constitue une entrave injustifiée à la liberté d'entreprendre et un dévoiement du statut salarial. À propos de dévoiement, le texte prévoit en outre comme seule échappatoire à un statut salarial forcé la coopérative d'activité et d'emploi.

de s'unir. Imposer cette forme sociale présenterait le danger de dévoyer le projet des coopératives d'activité et d'emploi et de leur faire perdre en pouvoir et en démocratie.

peut avoir des avantages : il introduit plus de concurrence dans des domaines qui en étaient parfois trop protégés et les consommateurs bénéficient, dans certains cas, de services de meilleure qualité à des prix plus compétitifs. cette nouvelle économie présente parfois une dimension plus sombre, une dimension où l'entrepreneur n'est entrepreneur que sur le papier, tandis que, dans les faits, il est sous la dépendance d'un client qui n'est autre que son donneur d'ordre. Le groupe Les Indépendants partage les préoccupations que soulève la situation d'une partie des entrepreneurs de la nouvelle économie. Nous observons en effet que certaines relations commerciales constituent en réalité des relations salariales, comme en témoignent plusieurs décisions de jurisprudence. La solution qui nous est proposée est simple, mais elle est peut-être trop simple. Il faudrait que tous les actifs rentrent dans la case du salarié ; à gauche, on propose l'entrepreneur salarié, encore plus à gauche, le salariat pur et simple, mais les situations des actifs sont parfois trop diverses pour correspondre à un seul statut. La présente proposition de loi consiste à rendre obligatoire, pour les travailleurs recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes numériques, d'être soit salariés de cette plateforme, soit entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi. Cette solution nous paraît problématique à plus d'un titre. D'abord, parce que la loi qui régit les coopératives dispose, en son article 1, que « La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies ». Ainsi, la création ou l'intégration d'une coopérative, comme de toute société, repose sur le consentement des intéressés. L'obligation, même proposée dans un but de protection des actifs concernés, nous semble contraire au principe de la coopérative. Une autre difficulté est soulevée par le périmètre de la proposition de loi que nous examinons : celui-ci ne concerne que les plateformes de mise en relation par voie électronique. Il nous semble que le problème posé par une relation commerciale qui dégénère en relation de dépendance, voire en salariat, est un problème plus large, qui ne peut être réduit à ces seules plateformes numériques. Enfin, cette solution viendrait alourdir un peu plus encore le marché de l'emploi. Les plateformes du numérique ont beaucoup de torts, mais il faut leur reconnaître qu'elles ont démontré à ceux qui en doutaient que le coût du travail salarié en France est un véritable frein à l'emploi. La protection sociale des travailleurs n'est évidemment pas une aberration à nos yeux. Pour nous, l'aberration est de conditionner la protection sociale au statut des individus. Nous souhaiterions voir l'émergence d'un système de protection sociale unifiée-

Un tel système ne saurait cependant s'imposer à ceux qui ne le souhaitent pas, lesquels devraient pouvoir rester libres de s'en affranchir et recourir à d'autres moyens de financement de leur protection sociale. Le problème soulevé par cette proposition de loi est aussi celui de la dépendance économique. En effet, ce que rencontrent les entrepreneurs individuels, les TPE et les PME le rencontrent aussi : ce sont les pratiques anticoncurrentielles, les abus de position dominante ou encore les ruptures brutales de relations commerciales. La très grande majorité des entreprises françaises sont des TPE et PME. Elles sont dynamiques, innovantes ; elles sont une chance pour notre pays. Cependant, elles sont, comme les auto-entrepreneurs, susceptibles de tomber sous le joug de la dépendance économique d'un donneur d'ordre. C'est à la puissance publique qu'il échoit de déterminer et de faire respecter les règles de la concurrence. Cette concurrence doit être loyale et effective, afin de refléter les intérêts de chacun des acteurs. C'est elle qui permet aux petits entrepreneurs de ne pas se retrouver en situation de dépendance économique. économique. La proposition de loi soulève donc un double problème : celui de la protection sociale des travailleurs et celui de la dépendance économique. Il n'est pas résolu en l'état actuel du présent texte, mais il faut reconnaître à celui-ci le mérite d'aborder les difficultés des petits entrepreneurs.

qui bouleverse le fondement même que nous lui connaissons actuellement. Nous constatons en effet une organisation plus déshumanisée, puisqu'elle est gérée et fondée sur des algorithmes, des taux de marge très faibles et une flexibilité des heures de travail très large. C'est pourquoi, consciente de ce nouveau schéma, la commission des affaires sociales a créé une mission d'information relative au « droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants ». Le 3 juillet 2019, le président Alain Milon nous nommait, Frédérique Puissat, Michel Forissier et moi-même, rapporteurs de cette mission. Nos travaux ont commencé en septembre dernier, et les conclusions doivent être rendues au printemps. Comme son nom l'indique, notre mission est amenée à étudier ce sujet dans son ensemble. Ce champ comprend notamment le droit du travail, le traitement social et la protection sociale des travailleurs concernés. Plus généralement, comme l'a dit mon collègue, cette mission pourrait être l'occasion d'une réflexion sur les enjeux actuels du statut d'indépendant.

une réflexion plus aboutie. Sur la forme, évalué à 1 % de la population active, le nombre exact de travailleurs est difficile à estimer : l'activité peut être totale, secondaire ou même d'appoint. est tout aussi complexe de connaître avec précision les rémunérations, puisque certains opèrent sur plusieurs plateformes. Les statistiques relatives aux travailleurs des plateformes sont difficiles à trouver et donc à exploiter. De plus, tous les modèles de plateformes ne sont pas comparables. D'une part, certaines plateformes se limitent à un rôle de mise en relation, sans influencer les coûts et les conditions de travail- c'est le cas de Malt. D'autres déterminent le prix, mais pas les conditions de travail, comme Brigad.

D'autre part, il apparaît important de préciser le modèle de développement des acteurs du numérique, notamment de ces plateformes. La spécificité majeure du modèle d'affaires des plateformes réside surtout dans l'effet réseau, qui les conduit à investir d'emblée des ressources importantes pour s'inscrire dans un contexte mondial exigeant. Les effets monopolistiques liés à cet effet réseau ne sont pas sans poser question, notamment quant à la soutenabilité de ce modèle économique particulier il amène les entreprises de l'économie numérique à faire des levées de fonds massives, alors que leurs investissements en « capital de production » sont très faibles par rapport à une entreprise classique. Il leur faut se développer rapidement, sans chercher de prime abord la rentabilité- elles ne considèrent que la croissance. En effet, quand le marché arrive à maturité, les plus gros rachètent les plus petits et se partagent le marché en situation de quasi-monopole. C'est le cas, actuellement, de moteurs de recherche ou de réseaux sociaux. Pour toutes ces raisons, la proposition que nous examinons aujourd'hui n'apporte pas une réponse suffisante. Tout n'est pas aussi simple, et le statut coopératif, tel qu'il est défini, paraît succinct. Sur le fond, cette proposition de loi appelle un certain nombre d'observations. Elle s'appliquerait à toutes les plateformes numériques, y compris celles dont le mode de fonctionnement ne pose aujourd'hui aucun problème. L'économie numérique constitue un enjeu important en termes d'économie future et de création d'emploi. Il convient de ne pas fragiliser un secteur qui permet à un certain nombre de nos concitoyens de sortir du chômage. Si les conditions de travail et de rémunération ne sont pas toujours satisfaisantes, c'est peut-être aussi lié à la situation de notre marché du travail. En effet, la situation des travailleurs des plateformes n'est pas nécessairement moins favorable que celle des salariés enchaînant des contrats très courts ou travaillant dans l'économie souterraine. Le salariat ne correspond pas nécessairement non plus aux aspirations de tous les travailleurs concernés. Nous avons constaté que, quelles que soient les activités exercées, c'est la recherche d'une liberté, d'une indépendance et d'une autonomie que ces travailleurs appréciaient : choix des horaires et des tarifs, travail sur plusieurs plateformes ... Force est de constater que la protection sociale n'est pas une priorité pour ces travailleurs, majoritairement jeunes et qui ne sont pas encore sensibilisés aux accidents de la vie, le sont que peu. Il nous appartient donc de travailler sur ce volet. Si la protection sociale des travailleurs des plateformes peut être améliorée, il convient plutôt de construire une protection sociale universelle et déconnectée du statut. La mission doit encore enrichir ses travaux par des auditions complémentaires et une étude comparative des expériences de nos voisins européens ou d'autres États, tels le Canada ou encore les États-Unis.

Vos travaux sont intéressants en termes d'alerte et de communication. Il est de notre responsabilité de parlementaires de nous en approprier. Cela dit, je rappelle que la commission des affaires sociales, en la personne de son président, Alain Milon, s'en était saisie bien en amont, dès la fin du mois de juin 2019. Je salue doublement cette démarche insistante et unanime des sénateurs, car je viens d'apprendre que Jean-Yves Frouin a été missionné par M. le Premier ministre sur le sujet proposition de loi apparaît incomplète. Le groupe Union Centriste vous propose donc de voter contre, mes chers collègues. L'objectif partagé avec la commission des affaires sociales est vraiment d'élargir la réflexion, dans le but d'aborder l'enjeu social et sociétal

Les plateformes numériques permettent aujourd'hui la mise en relation entre les travailleurs et des donneurs d'ordre. Il s'agit de prestations de différentes natures, dans de nombreux domaines d'activités. Le statut de micro-entrepreneur permet aux travailleurs de réaliser leurs missions dans le cadre d'une dépendance économique pouvant être considérée, dans certains cas, comme un lien de subordination. Le risque est grand de voir cette relation requalifiée en contrat de travail par les tribunaux. Cette fragilité juridique n'est pas satisfaisante. Se pose également la question de la répartition des profits et des garanties sociales pour ces travailleurs, qui, aujourd'hui, dans leur grande majorité, ne veulent pas être salariés ils souhaitent garder leur indépendance et avoir une activité modulable, éventuellement exercée parallèlement à un autre emploi ou à une autre fonction. À ce stade de nos travaux, nous constatons que la réalité de la situation des travailleurs indépendants économiquement dépendants des plateformes est hétérogène et représente encore une part marginale de la population active. En premier lieu, les plateformes numériques sont diverses. Un certain nombre de plateformes, correspondant à la définition de l'article 242 du code général des impôts, se bornent à un rôle de mise en relation entre des travailleurs indépendants et des clients. Ces plateformes n'interviennent ni pour fixer le prix des prestations ni pour organiser les conditions dans lesquelles ces prestations sont effectuées. On connaît, par ailleurs, des plateformes de services organisés hors ligne, qui fournissent des prestations standardisées délivrées par des professionnels, notamment dans les secteurs de la conduite de voitures de transport avec chauffeur et de la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues. Elles sont devenues, depuis quelques années, les plateformes les plus visibles et celles dont le développement soulève le plus de questions. Ces plateformes déterminent à la fois les caractéristiques de la prestation et son prix, notamment par le biais d'algorithmes, et apparaissent, de ce fait, comme les plus exposées au risque juridique de requalification en contrat de travail. Ainsi, si l'activité de conducteur de VTC s'est profondément professionnalisée, du fait notamment des coûts d'entrée représentés par l'obtention d'une licence et l'acquisition ou la location d'un véhicule, les services de livraison à vélo semblent plus souvent correspondre à une activité à la fois temporaire et secondaire pour les travailleurs concernés. On peut aussi citer les plateformes de micro-travail, qui consistent à l'externalisation de tâches fortement fragmentées et à faible valeur ajoutée. Le micro-travail représente une activité généralement très accessoire, le revenu mensuel moyen généré sur les plateformes concernées ne dépassant pas quelques dizaines d'euros. Ainsi, compte tenu de la diversité des activités, allant du job étudiant à la mise en relation de cadres de haut niveau travaillant en France, il est nécessaire de bien mesurer les impacts du cadre législatif sur l'ensemble des activités avant de légiférer. En deuxième lieu, les membres du groupe Les Républicains rappellent que les travailleurs des plateformes ne constituent pas une catégorie statistique en tant que telle et qu'il reste difficile d'estimer leur nombre avec précision. On parle de 100 000 personnes qui exerceraient leur activité exclusivement une plateforme, dont un quart de chauffeurs de VTC, ou de 200 000 personnes qui auraient recours à un intermédiaire pour l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il s'agisse ou non d'une plateforme numérique et que cette activité soit leur activité principale ou une activité d'appoint. En ce qui concerne la question de la protection sociale, il convient de rappeler que tous les travailleurs des plateformes bénéficient des protections universelles- santé, famille -et cotisent à l'assurance retraite. L'absence d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et d'assurance chômage est, en outre, propre au statut d'indépendant et doit être mise en relation avec l'absence de cotisation au titre de ces risques. Nous sommes attachés à ce que tous les travailleurs bénéficient d'une protection universelle,

Je me permets, à cette occasion, de vous rappeler que, lors de l'examen du texte par le Sénat, nous nous étions opposés au principe même de cette charte, en évoquant justement sa fragilité constitutionnelle. plateformes constitue, dans le cadre de l'économie numérique, un moyen de retour à l'emploi et une chance de sortir de la précarité pour un nombre non négligeable de chômeurs de longue durée relégués dans de petits boulots ou même dans l'économie souterraine. Les travailleurs concernés ne souhaitent pas devenir salariés- il faut le dire ! Ils sont attachés à leur indépendance et à leur autonomie dans leur travail. L'adhésion à une coopérative d'activité et d'emploi ne peut, à notre sens, être obligatoire. Cela serait contradictoire avec le principe de liberté d'entreprendre, que Les Républicains estiment fondamental dans notre choix de société. Nous considérons que les travaux et la réflexion engagée pour la préparation de cette proposition de loi sont des éléments à intégrer et constituent un apport pour notre mission d'information. Nous pouvons aussi penser qu'il s'agit, pour les auteurs, d'un texte d'appel. Nous sommes également convaincus de la nécessité de permettre à ce modèle économique d'exister, en raison de son utilité. Ce n'est pas en établissant un texte dans l'urgence que nous apporterons des solutions globales aux problèmes qui se posent ! Nous souhaitons aller au bout de la mission. Ensuite, nous pourrons engager, ensemble, une réflexion sur l'adaptation du cadre législatif, dans les principes de notre modèle social, qui qui doivent être respectés par tous les modèles économiques émergents. Pour conclure, je dirai que la proposition de loi présentée aujourd'hui ne peut apporter une solution viable et ne répond ni aux attentes exprimées par les travailleurs ni à celles des responsables des plateformes. Le groupe Les Républicains propose d'aborder de façon plus globale l'enjeu du développement de l'économie des plateformes numériques, en enrichissant le travail parlementaire des travaux de la mission d'information. Nous voterons, bien entendu, contre la proposition

de façon encore plus poussée que le recours à la sous-traitance « classique ». L'économie des plateformes, également appelée « économie collaborative » ou encore « ubérisation », recouvre des situations très diverses, mais connaît une forte croissance.

En termes de politiques publiques, en particulier de droit du travail, l'économie des plateformes prolonge les questionnements sur la diversification des formes d'emploi, avec l'idée d'un statut intermédiaire entre salarié et travailleur indépendant classiques, sur la sécurisation des parcours professionnels et, enfin, sur l'adaptation du système de prélèvements obligatoires. L'article 60 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou « loi El Khomri », a créé au nouveau titre dans le code du travail, relatif aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. L'article L. 7341-1 en définit ainsi le champ d'application Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 du code général des impôts. Ce titre clarifiait les obligations sociales des plateformes en ligne et précisait les droits des travailleurs concernés en matière d'accidents du travail, de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience et de droit syndical. Ces dispositions, qui accordaient quelques droits sociaux aux travailleurs indépendants travaillant sur des plateformes collaboratives, en leur faisant bénéficier de certains attributs du salariat, sans toutefois que ces éléments soient, d'une quelconque façon, de nature de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, avaient été introduites lors de l'examen parlementaire, en commission, à l'Assemblée nationale. Elles avaient été supprimées par le Sénat par un amendement des corapporteurs, dont mon prédécesseur à cette tribune et moi-même. nous avions alors jugé ces dispositions prématurées, notamment au regard des affaires juridictionnelles en cours au moment de l'examen du projet de loi, tendant à requalifier certains contrats de travailleurs de plateformes en contrats de travail salarié. Lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ces dispositions furent rétablies, avec, toutefois, une modification substantielle, répondant à la critique formulée par les corapporteurs du Sénat sur l'ambiguïté de l'article créant, dans le code du travail, un statut de travailleurs non salariés sans être indépendants, la disposition selon laquelle la reconnaissance de la responsabilité sociale de la plateforme à l'égard de ces travailleurs n'entraînait pas de lien de subordination.

collègues, vous avez raison de vous interroger sur la nature du contrat et des relations entre les plateformes et les travailleurs dits « indépendants ». Il y a bien lieu d'élaborer un statut spécifique d'indépendant, d'encadrer les relations contractuelles avec les plateformes et, peut-être, d'encourager la création d'une branche professionnelle qui permettra de définir des droits concrets. En revanche, la réponse que vous apportez avec cette proposition de loi ne peut constituer qu'une solution parmi d'autres. Elle ne saurait répondre à l'ensemble des situations et pourrait même ne pas convenir à certains indépendants.

Les travailleurs des plateformes représentent 200 000 personnes en France, soit 0,8 % des actifs occupés. Parmi ceux-ci, nous pouvons distinguer trois catégories de travailleurs : ceux qui sont salariés et utilisent les plateformes afin de compléter leurs revenus, ceux qui sont travailleurs indépendants et utilisent les plateformes comme forme d'activité exclusive et ceux qui sont hautement qualifiés et souhaitent bénéficier de davantage de flexibilité en se tournant vers un intermédiaire numérique, comme les. La première de ces catégories est couverte par la protection sociale des salariés. En revanche, les deux autres font l'objet de débats. Actuellement, la loi prévoit des droits individuels, tels que la prise en charge, plafonnée par décret, de la cotisation du travailleur pour une assurance couvrant le risque d'accidents du travail, un droit d'accès à la formation professionnelle continue et le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience, et des droits collectifs, tels que la protection des travailleurs participant à des mouvements en vue de la défense de leurs revendications professionnelles ou encore la faculté pour les travailleurs visés de constituer une organisation syndicale. En outre, le Gouvernement a souhaité approfondir cette démarche de régulation de la relation entre plateformes numériques et travailleurs indépendants au travers du projet de loi d'orientation des mobilités, notamment à l'article 20 Déposée le 28 novembre 2019 par des sénateurs du groupe socialiste et républicain, la présente proposition de loi part du postulat que les plateformes de mise en relation par voie électronique précarisent les travailleurs et « utilisent des algorithmes favorisant l'effacement des avancées sociales du siècle dernier », menaçant ainsi la « citoyenneté sociale » et la « solidarité nationale Afin de réguler la relation entre les travailleurs numériques et les plateformes, les auteurs de cette proposition de loi proposent d'obliger les travailleurs qui recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique sans en être salariés à être des entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi. Ainsi leur activité s'inscrirait dans le cadre juridique existant, à l'instar du statut d'entrepreneur salarié en CDI. Si l'objectif est louable, de nombreuses réserves ont émergé en commission des affaires sociales, pour plusieurs motifs, auxquels nous souscrivons. Il est difficile de contraindre l'ensemble de ces travailleurs à créer des coopératives d'activités et d'emplois, en raison souvent de leurs aspirations, tournées vers une recherche de liberté, d'indépendance et d'autonomie. La diversité des plateformes n'est pas prise en compte. En effet, la notion de « plateforme » recouvre une grande diversité d'acteurs. Les conditions des travailleurs sont aussi diverses que les plateformes elles-mêmes et ne sont pas forcément plus mauvaises que celles des salariés d'une CAE. Par ailleurs, comme je l'ai expliqué précédemment, la loi d'orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, autorise, à travers son article 20 et dans un délai d'un an, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. Enfin, la commission des affaires sociales a lancé, en septembre 2019, une mission d'information sur le droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants. Il est essentiel, selon nous, d'attendre les conclusions de ce rapport.

nous ne disons pas que notre proposition est la solution unique et miracle. Comme certains l'ont dit, elle permet d'ouvrir le débat à des alternatives diverses, visant à mieux protéger les travailleurs plutôt qu'à tenter de protéger les plateformes. C'est le sens de notre solution des coopératives d'activité et d'emploi, dites « CAE

il n'existe que depuis 2014. Il a été conçu comme une alternative à l'auto-entrepreneuriat. Je comprends donc que certains prennent leurs distances à l'égard de cette proposition.

pour améliorer la situation de ces travailleurs exploités, pour leur dire et leur faire comprendre que nous les entendons et que nous les défendons. Je veux saluer ici tous ces travailleurs qui se mobilisent individuellement : ce sont de véritables lanceurs d'alerte, respect ! Le débat que nous tenons aujourd'hui est une étape importante et nécessaire dans la construction de la protection sociale à la française du XXI siècle, forte de son histoire, solide sur ses fondamentaux et adaptée aux évolutions du monde. En adoptant cette proposition de loi, vous permettrez à nos collègues députés de se saisir de ce débat et d'entamer la construction de cet édifice. Comme l'écrivait Goethe : « On peut aussi construire quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin ». La discussion La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l'article

Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.